c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre collègue Alain Bertrand. Il luttait avec courage, depuis plusieurs mois- nous le savions -, contre une grave maladie. Il s'est éteint ce matin à l'hôpital de sa ville de Mende. Il était sénateur de la Lozère depuis 2011.

il devient vice-président du conseil régional en 2004 et le reste jusqu'en 2011. Il est élu maire de Mende en 2008, puis sénateur du département de la Lozère en 2011. Au sein de notre assemblée, il fut un défenseur acharné des territoires ruraux, et même des territoires « hyper-ruraux

de même qu'il ne peut y avoir de sous-citoyen et de minorité sacrifiée et interdite d'avenir », il appelait dans ce rapport les habitants et les acteurs de l'hyper-ruralité à « ne pas baisser les bras, à se mobiliser, individuellement ou collectivement », pour s'opposer à cette « fatalité qui n'en est pas une » et faire de ces territoires trop souvent oubliés un atout pour notre pays. Ceux qui l'ont côtoyé se rappellent un homme affable, chaleureux, plein d'humour. Au nom du Sénat, je souhaite exprimer notre sympathie et notre profonde compassion à sa famille, à ses proches, ainsi qu'au président et aux membres de son groupe, le RDSE. Je vous propose d'observer un instant de recueillement en sa mémoire.

madame le ministre, mes chers collègues, pardonnez-moi : c'est le jour des mauvaises nouvelles -, c'est avec émotion et tristesse que nous avons appris la disparition de notre ancien collègue Michel Charasse, qui nous a quittés le 21 février dernier à l'issue d'un combat très courageux contre une cruelle maladie. Nous nous étions revus récemment encore, en janvier de cette année, lorsque le Président de la République lui avait remis les insignes d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, ordre dans lequel je l'avais moi-même reçu en 2011- je l'avais décrit alors comme un « républicain absolu J'étais présent, avec vous, madame la garde des sceaux, et avec nos collègues du département du Puy-de-Dôme, à la cérémonie d'adieu organisée mercredi dernier à Puy-Guillaume, à laquelle ont assisté de nombreuses personnalités. Figure de notre vie politique, Michel Charasse était un serviteur passionné de la République, qui constituait pour lui la référence essentielle et dont il prônait inlassablement les valeurs. C'est autour de ses indéfectibles convictions républicaines que se sont articulés tous les grands engagements de sa vie publique, comme élu local, comme conseiller du Président de la République François Mitterrand, comme ministre, comme sénateur ou comme juge constitutionnel. Profondément attaché à la liberté individuelle, et tout particulièrement à la liberté de conscience, c'était un défenseur intransigeant de la laïcité. Les règles républicaines devaient selon lui s'appliquer d'une manière égale à tous, sans distinction d'origine, de croyances, d'intérêts ou de communautés, uniformément sur le territoire de la République, une et indivisible. La fraternité s'incarnait chez lui par une grande fidélité en amitié et une générosité qui s'illustra notamment par son soutien constant aux Restos du coeur. Sa forte personnalité, parfois atypique, souvent truculente, sa passion pour la chasse et les moments de convivialité attablés, son indépendance d'esprit, sa liberté de parole, sa cohérence et sa détermination dans l'expression de ses opinions, son humour parfois provocateur ont laissé un souvenir marquant et durable dans notre assemblée, où il siégea pendant nombre d'années. C'était aussi un travailleur acharné, qui fit bénéficier le Sénat de ses compétences de fin juriste et de son expérience du monde parlementaire. Il était né le 8 juillet 1941 à Chamalières, dans le département du Puy-de-Dôme, auquel il restera toujours fidèle, d'une mère corse et d'un père auvergnat, tous deux salariés de la Banque de France et militants syndicaux. Titulaire d'une licence en droit et d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, il commença sa carrière au service de l'État comme attaché d'administration centrale au ministère de l'économie et des finances. Engagé en politique dès l'âge de 21 ans, par son adhésion à la SFIO, il s'immergea très vite dans le monde parlementaire en travaillant à l'Assemblée nationale comme assistant de plusieurs députés, puis comme secrétaire général adjoint du groupe socialiste, où il devint un expert du droit constitutionnel, de la procédure parlementaire et des finances publiques. Après un premier et bref mandat électoral en Corse, Michel Charasse fut élu maire de Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme, en 1977.

En 1981, Michel Charasse fit son entrée au Sénat ; il remplaçait Roger Quilliot, devenu ministre. Réélu sénateur en 1992 et en 2001, il ne quittera plus notre assemblée jusqu'à sa nomination au Conseil constitutionnel en 2010, hormis, bien sûr, les quatre années où il exerça des fonctions ministérielles, entre 1988 et 1992. De 1981 à 1995, parallèlement à ses fonctions de sénateur, il fut aussi et surtout un très proche et confiant conseiller du Président de la République. Alors installé à l'Élysée, où il passait la majeure partie de son temps, il fit preuve jusqu'au bout d'une fidélité et d'un dévouement sans faille envers le Président Mitterrand. Ministre chargé du budget de 1988 à 1992, Michel Charasse fut l'un des titulaires les plus endurants de ce poste exposé. Son passage y fut notamment marqué par le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, la normalisation de l'imposition des élus ou encore la modernisation de la fiscalité locale.

Il fut un membre éminent, assidu et écouté, de notre commission des finances, où il s'illustra tout particulièrement comme rapporteur spécial des crédits de l'aide au développement. Il conféra toute sa portée aux prérogatives de contrôle « sur pièces et sur place », en effectuant un certain nombre de missions à l'étranger, notamment en Afrique, dont il était devenu un grand connaisseur. Après avoir été secrétaire du Sénat de 1995 à 1998, puis membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes, Michel Charasse exerça, de 2001 à 2004, l'importante responsabilité de questeur du Sénat du Sénat ; dans ce cadre, il se montra un gardien très attentif de l'autonomie de notre assemblée. En 1999, il joua par ailleurs un rôle marquant au sein de la commission d'enquête sénatoriale sur la conduite de la politique de sécurité menée par l'État en Corse. Au long de ses mandats sénatoriaux, il se distingua en outre par ses prises de position affirmées sur les questions concernant la justice et les relations avec les juges, notamment en faveur du maintien des liens entre la Chancellerie et le parquet, ou en faisant valoir l'immunité parlementaire pour refuser de déférer à des convocations adressées par des juges- nous en avons quelques souvenirs. Attaché au bicamérisme, Michel Charasse se plaisait à souligner l'excellence du travail législatif du Sénat, considérant que « Les textes qui sortent de cette maison sont imprégnés de bon sens et de [la] pratique du terrain ». En 2010, Michel Charasse, reconnu depuis longtemps comme un grand spécialiste du droit constitutionnel, fut nommé membre du Conseil constitutionnel par le Président de la République Nicolas Sarkozy. Il déclarait alors, dans un entretien au : « Je suis un homme libre et indépendant, qui sert la République, qui sert ses institutions et veut les préserver dans ce qu'elles ont de plus fondamental pour l'équilibre de la France. »

je souhaite rendre aujourd'hui un hommage solennel à un grand serviteur de l'État, à un grand républicain, à une figure marquante de notre vie politique et parlementaire. À son épouse Danièle, à ceux qui ont partagé ses engagements, je souhaite redire la part que le Sénat prend à leur deuil. Michel Charasse était une figure qui restera présente dans cet hémicycle.

Mes chers collègues, L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (projet n° 283, texte de la commission

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, au milieu de sujets de préoccupation plus importants, et après deux hommages empreints d'émotion, nous avons à nous prononcer sur plusieurs questions : le Parquet européen, des compléments concernant le PNAT une juridiction spécialisée en matière d'environnement, l'extension des conventions judiciaires dites d'intérêt public, ainsi que diverses mesures, dont trois sont particulièrement susceptibles de retenir votre attention. du Parquet européen, saluons sa création et apprécions son organisation. Vous saluerez sa création si vous croyez à la construction à la construction européenne, si vous pensez qu'on lutte mieux à l'échelle de l'Union européenne contre les atteintes aux intérêts financiers de l'Union, c'est-à-dire, concrètement, contre la corruption et la fraude transfrontalière à la TVA, si vous êtes convaincu que l'Europe n'est pas simplement un marché unique ou une monnaie, mais qu'elle est aussi un État de droit, et que cela a du sens dans un monde qui ne croit plus qu'aux rapports de force. Vous saluerez son organisation si vous êtes attentif à la souveraineté nationale, en particulier à notre souveraineté judiciaire. Il comportera deux niveaux

pragmatique, propre, pour un Parquet européen que nous espérons opérationnel à la fin de l'année. Deuxième volet : le parquet national antiterroriste et le parquet national financier. avec l'accord de tous les professionnels, le rôle du PNAT en matière d'entraide judiciaire et étendrez sa compétence aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation- il s'agit essentiellement des affaires d'espionnage,

Sur proposition du procureur général Molins, vous apporterez la dernière pierre à notre système de résolution des conflits entre juridictions. J'en viens aux juridictions spécialisées.

Ce n'est pas une juridiction nouvelle qui vous est proposée, simplement une juridiction qui connaîtrait d'un peu plus de dossiers et serait, à ce titre, sinon spécialisée, du moins un peu plus spécialisée.

la convention judiciaire d'intérêt public au domaine de l'environnement. Cette convention judiciaire d'intérêt public, vous la connaissez bien, depuis la loi Sapin. Vous avez pu

en prévoyant un solide garde-fou en termes de libertés publiques, l'adaptation de la peine prononcée par le juge aux impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale.

vous donnerez sa conclusion à un débat qui a opposé ceux qui pensent qu'il faut laisser les professions se gérer elles-mêmes et ceux qui pensent, à l'inverse, que l'entre soi n'est pas bon dans la durée. La commission des lois a essayé de trouver un équilibre

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer cet après-midi constitue la dernière étape sur la voie de ce que le Conseil d'État avait qualifié en 2011 de « saut qualitatif majeur » pour la coopération judiciaire européenne. Le Parquet européen, créé en 2017 par 22 États membres après de longues années de discussion, nécessitait en effet une adaptation de l'ordre juridique national pour pouvoir être pleinement opérationnel. C'est ce à quoi s'attache le présent projet de loi, qui permettra à cette nouvelle instance de s'attaquer, dès la fin de cette année, aux diverses infractions pénales portant préjudice aux intérêts financiers de l'Union européenne, c'est-à-dire à celles qui affectent soit la perception de ses recettes issues de la TVA et des droits de douane, soit l'exécution de ses programmes de dépenses comme les fonds structurels ou les aides de la PAC. En effet, si le marché unique est un acquis fondamental qui a permis d'élargir considérablement le champ d'action de nos entreprises, force est de constater qu'il a également élargi celui des fraudeurs. Ainsi la fraude transfrontalière à la TVA, très largement pratiquée par des groupes criminels organisés, a-t-elle progressivement atteint des proportions colossales ; elle représenterait chaque année plus de 50 milliards d'euros. Malgré leurs mérites réels, Eurojust, Europol ou l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) n'ont pas permis d'endiguer ce phénomène, notamment parce qu'ils ne disposent pas des prérogatives nécessaires. le Parquet européen, lui, les aura : il pourra diligenter des enquêtes dans plusieurs États membres, engager lui-même des poursuites et faire accepter par n'importe quelle juridiction nationale les éléments de preuves qu'il recueillera. Il ne sera pas pour autant l'organe excessivement centralisé qu'avait initialement imaginé la Commission européenne. Grâce à l'action du Sénat et de treize autres parlements nationaux pour faire respecter le principe de subsidiarité, le Parquet européen sera organisé selon deux axes clés. La collégialité, d'une part, assurera la participation d'un représentant de chaque parquet national à la définition de sa politique pénale ; la décentralisation, permettra son ancrage dans les structures et l'ordre juridiques de chaque État membre. Cette solution est à la fois plus équilibrée et plus respectueuse de la souveraineté nationale. Elle ne doit toutefois pas nous conduire à ignorer le défi que représentera l'articulation opérationnelle de cette construction inédite avec les juridictions françaises. Le dispositif mis en place, notamment autour des prérogatives du procureur européen délégué, vient en effet bousculer, rien de moins, l'ordonnancement traditionnel de notre cadre procédural. La commission des lois, cher président Bas, a apporté des précisions utiles en la matière, mais celles-ci ne rendront pas moins nécessaire l'observation attentive de la façon dont le Parquet européen exercera ses missions dans notre pays. Le pragmatisme nous invite donc à examiner d'abord, dans les années à venir, son efficacité et sa plus-value, ainsi que son insertion harmonieuse dans le cadre des justices nationales, avant de songer à étendre ses compétences, comme ont d'ores et déjà pu en émettre le souhait la Commission européenne ou le Président de la République française. Alors que le Parquet européen n'a même pas encore commencé ses travaux, un tel appel est pour le moins prématuré. Dans l'immédiat, je crois plus utile de se concentrer avant tout sur la réussite de cette initiative visant au développement d'une Europe capable de mieux protéger ses intérêts et de lutter plus efficacement contre la délinquance financière. Très bien ! J'en viens aux dispositions du projet de loi relatives à la justice pénale spécialisée. Ce texte a permis au Gouvernement d'inscrire dans la loi plusieurs précisions techniques qui étaient attendues et nécessaires. Ainsi en est-il des articles portant sur le règlement des conflits de compétences entre juridictions spécialisées et non spécialisées ou sur l'élargissement des compétences du parquet national antiterroriste et du parquet national financier, parquet national financier, autant de dispositions cohérentes auxquelles notre groupe souscrit. En revanche, l'introduction dans le projet de loi de dispositions relatives aux instructions générales des parquets en matière de direction d'enquête est plus surprenante elle révèle le caractère à tout le moins fourre-tout- il faut le dire -du texte qui nous a été soumis. Il était certes primordial de revenir sur l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 décembre dernier, qui soulevait des difficultés pratiques considérables, en imposant aux enquêteurs et aux procureurs des exigences formalistes chronophages. Je me permets néanmoins, à titre personnel, de m'interroger sur le lien entre ce dispositif et le Parquet européen ou encore la justice spécialisée. En ce qui concerne le volet ayant trait à la justice environnementale, je me limiterai à de brèves observations. Si l'instauration de la convention judiciaire d'intérêt public permettra certainement de rendre plus efficace la répression des atteintes à l'environnement, il sera essentiel que les services compétents du ministère de l'environnement contrôlent la réalité de la régularisation de la situation de la personne morale partie à la convention et l'effectivité de la réparation du dommage écologique. En revanche, le caractère rare et complexe d'un contentieux ne justifie pas à lui seul la création de pôles spécialisés. De plus, l'efficacité d'une politique pénale ne repose pas seulement sur la spécialisation de magistrats. Il est donc à craindre que l'instauration des pôles de justice environnementale n'améliore pas significativement l'efficacité de la politique pénale en la matière, sinon qu'elle ajoute de la complexité à l'organisation judiciaire et à sa lisibilité. permettez-moi de me satisfaire de l'adoption de l'amendement que j'avais déposé, et que mes collègues ont bien voulu adopter, relatif à la création de nouveaux offices par les professions juridiques réglementées. Merci, monsieur le président ! Mes chers collègues, pour l'ensemble des raisons évoquées, je ne doute pas qu'un nombre important des membres du groupe Les Républicains, si ce n'est leur totalité, apportera son soutien au présent projet de loi. Très bien ! La parole

devient trop souvent l'habitude et nous en payons les conséquences à chaque texte étudié si vite. Dans le cas présent, ce sont des avis pris à la va-vite sur des amendements. Des avis discutables et discutés Je ne comprends pas, par exemple, qu'un amendement soutenu par le Gouvernement et voté à l'unanimité ici puisse obtenir un avis défavorable quelques semaines après avoir été adopté dans un autre texte, en l'espèce celui qui avait été présenté par notre collègue Jérôme Tel a pourtant été le cas concernant un amendement visant à punir les atterrissages sauvages d'avions au sommet du Mont-Blanc. Le symbole est d'autant plus étonnant que l'on parle du lieu retenu par le Président de la République pour incarner son prétendu virage écologique. que ce n'est pas le fait que ce virage soit remis en question par de nombreux observateurs qui a pu amener le Gouvernement à rejeter un amendement qu'il a pourtant lui-même coécrit ! Mais j'imagine, madame la ministre, que vous aurez à coeur de nous rassurer. Au-delà de ces réserves de forme, maintes fois répétées et qui se veulent pédagogiques pour le Gouvernement, le groupe socialiste et républicain adoptera une position constructive sur ce projet de loi. En ce qui concerne le contenu relatif au Parquet européen, nous sommes convaincus et approuvons ce dispositif visant à mettre en place un règlement européen que nous soutenons. Nous n'avons pas relevé de difficulté majeure dans le schéma qui nous est proposé. Il vient conclure en quelque sorte le soutien de la France- un soutien actif, constant et de longue date -à la mise en place du Parquet européen, un combat de longue haleine dont nous nous félicitons et auquel nous avons pris part. Si toutes les interrogations sur l'indépendance du Parquet sur le territoire national ne sont pas levées, cela inspirera peut-être une évolution à venir. L'essentiel réside toutefois dans l'avènement consensuel de ce Parquet européen, qui contribuera à rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Nous avons eu, en revanche, des débats plus tourmentés sur les mesures environnementales de ce texte. Les premiers éléments constitutifs d'une justice spécialisée que vous nous avez présentés, madame la garde des sceaux, semblent résolument manquer d'ambition. L'instauration de pôles régionaux laisse sceptiques une grande partie des acteurs quotidiens de la justice, qui réclament surtout une hausse des moyens. Comme l'a relevé mon collègue Jacques Bigot, « il n'y a pas de poursuites de la part d'un procureur sans enquête ni dossier des agents chargés de l'environnement et de la constatation des délits. C'est vrai, aujourd'hui, devant les juridictions ordinaires de première instance. Ce sera vrai également, demain, devant ces nouvelles juridictions Mais le point de friction le plus notable réside dans la mise en place de la convention judiciaire écologique. Souvent présentée comme un progrès considérable par ses laudateurs, avec parfois force arguments dithyrambiques, elle permettrait de désengorger la justice et de garantir une réponse rapide aux infractions environnementales. Si le fameux « plaider-coupable » commence à entrer dans les moeurs dans certains secteurs, il ne saurait constituer une solution acceptable en matière environnementale. Et pourquoi ? Nous connaissons bien ce dispositif grâce aux apports de la loi Sapin II. Une entreprise qui fait de l'évasion fiscale crée un manque à gagner pour la collectivité. C'est grave, mais réparable, et la convention permet souvent de gagner en efficacité et en rapidité. Il faut relever que beaucoup ne font pas de cette solution une recette miracle ; je pense à certains collègues d'autres groupes. Mais il y a une différence flagrante avec une entreprise qui détruit notre environnement. Dans un tel cas, les dégâts provoqués sont bien souvent irrémédiables, comme vous l'avez vous-même fait remarquer en séance, madame la ministre. Pourquoi la société, si prompte d'ailleurs à réclamer durcissement des peines et exemplarité des sanctions en matière de justice, tolérerait-elle un tel laissez-faire en matière environnementale ? Toutes choses égales par ailleurs, pensez-vous que la marée noire de l'ou encore l'explosion de Lubrizol pourraient être réglées par une convention judiciaire ? Jusqu'où devons-nous encourager cette logique transactionnelle qui pointe son nez en matière de justice environnementale ? L'absence de procès dans les affaires réglées par convention aura par ailleurs bien d'autres conséquences, comme l'a rappelé François Molins, pour qui « il y a une vraie valeur pédagogique du procès et des débats qui peuvent se produire devant une juridiction pénale Nous sommes donc déçus par les aspects environnementaux contenus dans ce texte. Nous avons hésité quant aux conclusions à en tirer sur notre vote final. Nous conservons l'espoir que la Convention citoyenne pour le climat vienne améliorer les réponses existantes en matière de justice environnementale, puisque le Président de la République s'est engagé à en reprendre les conclusions sans filtre. Notre conservatisme parlementaire sera peut-être débordé par l'ambition de citoyens tirés au sort qui ont décidé de mener leur tâche avec détermination. L'instauration du crime d'écocide, par exemple, rejetée jusqu'ici au Sénat et à l'Assemblée nationale, pourrait ainsi nous être soumise de nouveau grâce à l'implication de citoyens débarrassés de tout Attendons Attendons ... Nous relevons cependant avec satisfaction l'adoption d'un amendement visant à permettre l'immobilisationd'un navire qui a jeté ses eaux de ballast dans les eaux territoriales, dans l'attente du paiement d'un cautionnement.

notamment l'article 8, mais avec une très grande conviction sur le Parquet européen. La parole

Bien sûr, après la sortie officielle et définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne le 1 février dernier, l'annonce d'une nouvelle coopération renforcée est une bonne nouvelle pour les partisans de l'Europe et d'une solidarité européenne efficace que nous sommes. Il faut aussi saluer les bonnes nouvelles bruxelloises qui parviennent jusqu'à Paris. L'introduction du procureur européen délégué dans notre procédure pénale rouvre en outre le débat franco-français sur le fonctionnement de nos juridictions pénales, qui a émergé à l'occasion de l'affaire d'Outreau. Faut-il maintenir un système dual ? Envisager la suppression du juge d'instruction ? Et renforcer, le cas échéant, les contre-pouvoirs face au procureur ? Dans cette mouture en effet, les droits de la défense face au procureur européen ont été adaptés en conséquence. l'examen de ce texte semble avoir ouvert plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Certes, le titre II permet des ajustements sûrement bienvenus après la création en urgence des parquets nationaux financier et antiterroriste. Et le titre III permet de maintenir des dispositifs remis en cause par des décisions du Conseil constitutionnel. Ces ajustements doivent cependant nous conduire à repenser la manière de légiférer dans une matière régalienne comme la justice. Ces dernières décennies, plusieurs réformes ont été décidées dans l'urgence, en réaction à des crises majeures- affaire Cahuzac, attentats -, et l'on se trouve aujourd'hui obligé de remettre la main à l'ouvrage pour consolider des dispositions écrites très rapidement. Les réformes de la justice n'échappent pas à la procédure accélérée, ce nouveau texte en est une fois de plus l'exemple. En parallèle, des questions fondamentales n'ont toujours pas été tranchées je viens de parler des équilibres institutionnels au sein des juridictions pénales et de la réforme de l'indépendance du parquet qui n'a toujours pas eu lieu. De même, la spécialisation des juridictions pose un problème d'accès à la justice, alors même que la carte judiciaire a été réformée pour être adaptée à la réorganisation territoriale. Soyons vigilants à rester totalement cohérents, et à ne pas renforcer les déséquilibres qui fragmentent déjà le territoire français en poursuivant la concentration administrative en région parisienne. Il faut enfin évoquer la question de la justice environnementale, un sujet qui prend de l'ampleur et qui mobilisera de plus en plus de magistrats dans les années à venir. Lorsque ces conflits ne sont pas pris en charge par nos tribunaux, ils s'expriment dans la violence et la provocation, parfois même dans l'illégalité.

C'est pourquoi nous espérons que la navette parlementaire permettra de renforcer les outils des juridictions, sur la base des nombreuses pistes proposées par notre groupe, en particulier par notre collègue Joël Labbé. Certaines dispositions du titre III, enfin, ne se rattachent ni à l'objectif d'instauration d'un Parquet européen ni au renforcement des juridictions spécialisées. De ce point de vue, elles ne nous semblent pas avoir leur place dans le texte aujourd'hui en discussion. En conclusion, la grande majorité de mon groupe votera ce texte, tandis que quelques-uns s'abstiendront au regard des réserves que j'ai exprimées en leur nom.

Il adapte tout d'abord la procédure pénale de notre pays à la mise en place en novembre prochain, à Luxembourg, de la nouvelle autorité judiciaire que représente le Parquet européen. Celui-ci sera compétent pour poursuivre les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, dont on estime, chaque année, le préjudice à plusieurs dizaines de milliards d'euros. La coopération renforcée, qui est instituée par ce texte dans le domaine judiciaire, correspond à une demande ancienne que notre pays a lui-même impulsée et que le Sénat a ardemment défendue dans les modalités qui ont été retenues. Cette partie du texte, plutôt consensuelle, a pu faire naître des inquiétudes quant à l'éventualité d'une disparition du juge d'instruction dans notre droit interne ou à l'ambivalence statutaire et l'indépendance du parquet. J'avais moi-même posé la question du modèle procédural applicable dans le cadre de la mise en place de ce Parquet européen. Ces doutes et inquiétudes ont été levés et, en tout état de cause, la pratique nous révélera rapidement ses premiers enseignements. Par ailleurs, ce texte renforce la justice pénale spécialisée, en particulier en matière d'atteintes environnementales. Pour ce dernier type de contentieux, on relève que les poursuites sont rares et les sanctions trop légères : seules 1 % des condamnations au pénal concerneraient l'environnement. C'est pourquoi la création d'une juridiction spécialisée au sein de chacune des trente-six cours d'appel, avec des magistrats dédiés, devrait permettre de rendre des décisions plus rapides et plus efficaces. La réponse pénale adaptée que le projet de loi met également en place par la voie d'une convention judiciaire d'intérêt public- la convention judiciaire environnementale -permettra d'obtenir une sanction plus rapide par le paiement d'une amende, d'une remise en état et, si celle-ci est impossible, d'une réparation du préjudice subi. Ces conventions, créées par la loi Sapin II, ont déjà fait leurs preuves en matière fiscale. Il ne fait aucun doute que la rapidité avec laquelle la sanction sera rendue, laquelle peut s'élever jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise mise en cause, conjuguée à la possibilité de rendre publique cette convention, sera de nature à rendre dissuasifs ces délits. Je me réjouis également que notre assemblée ait adopté des amendements permettant l'immobilisation d'un navire qui aurait jeté ses eaux de ballast dans les eaux territoriales, en attendant un cautionnement qui garantirait le paiement des amendes et la réparation des dommages. Cette nouvelle justice pour l'environnement que le Gouvernement met en place va bien évidemment dans le bon sens, même si malheureusement elle ne suffira pas aujourd'hui, à l'aune des scandales environnementaux qui ont fait l'actualité planétaire, à lutter contre la criminalité environnementale. C'est pourquoi il me semble urgent d'engager des discussions à l'échelle mondiale afin qu'une réglementation internationale voie enfin le jour. Pour conclure, le groupe La République En Marche ne peut que soutenir cette évolution majeure de la coopération européenne que représente le Parquet européen et l'adaptation du droit national à cette nouvelle institution européenne. Mon groupe approuve également le renforcement des juridictions pénales spécialisées, dont l'objectif est assurément de raccourcir les délais et d'apporter une plus grande maîtrise de la technicité du droit applicable.

ce projet de loi donne une grande place à la problématique de l'environnement, et il faut s'en réjouir. Il convient aussi de considérer que l'environnement est un domaine à la mode. Bien évidemment, on en rajoute, en oubliant parfois d'autres dossiers et domaines qui présentent un intérêt. Pour ma part, je me félicite des mesures très restrictives

contre la pollution créée par les rejets de fumées nocives par les grands navires qui consomment un fioul absolument horrible pour l'environnement. Sur ce point, l'Europe devrait faire quelque chose.

avec l'Irlande et les Pays-Bas, on peut faire le même constat. Ce n'est pas en créant un procureur européen ou un Parquet européen que l'on va régler cette difficulté. Il y a là une véritable problématique ! Il faut d'abord,

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il aura suffi d'une demi-journée pour boucler l'examen en séance de ce projet de loi aux dispositions aussi techniques que disparates moitié moins que ce qui était prévu, et bien moins encore que ce qu'auraient mérité de telles mesures. Il faut dire que la matière d'un tel projet ne se prêtait pas vraiment à un exercice conjoint d'écriture, le législateur étant invité à valider la loi plutôt qu'à participer à son élaboration. En ce qui concerne les dispositifs d'adaptation de notre droit national au Parquet européen, ceux-ci ont été construits au terme d'une dizaine d'années d'échanges entre l'Union européenne et ses États membres, parmi lesquels notre pays a été force de proposition, emmené par notre Haute Assemblée. Sur le fond, nous y sommes plutôt favorables, dans la version collégiale qui en résulte, même si l'assurance du rapporteur et de la garde des sceaux n'ont pas fini de nous convaincre sur les questions d'inamovibilité des magistrats français qui seront détachés pour endosser les fonctions de procureur européen Nous restons dubitatifs sur ce point, comme sur celui de la procédure « inventée » pour s'adapter à ce Parquet européen. Les États membres sont d'ailleurs plutôt issus d'une tradition inquisitoire, contrairement à notre pays qui suit un modèle accusatoire. Cela peut laisser craindre, comme l'a formulé le Syndicat de la magistrature, les « premiers pas vers la suppression du juge d'instruction ». Autre inquiétude pour l'avenir de ce Parquet européen : alors qu'il est, dans ses fondements actuels, cantonné aux affaires financières, il y a fort à craindre que son champ de compétences ne soit étendu dans les années à venir. Une fois l'édifice dressé, il semblera assez aisé, après son entrée en fonctions le 20 novembre 2020, d'y introduire, sous l'impulsion de l'Union européenne, de nouveaux champs. Je pense en particulier à la politique antiterroriste. Cela poserait alors un certain nombre de difficultés en matière de subsidiarité et de souveraineté, surtout

que ce Parquet européen reste concentré et aussi efficace que possible dans le cadre décidé : escroqueries à la TVA, faits de corruption, détournement de fonds publics, abus de confiance, blanchiment d'argent et certains délits douaniers. Il y a déjà fort à faire, et la manne financière à récupérer serait de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards pour la France ! Il y a donc du boulot En ce qui concerne les mesures de justice environnementale, nous sommes en revanche beaucoup plus dubitatifs sur les dispositifs proposés. Nous avons défendu la suppression de la convention judiciaire d'intérêt public en raison de son insuffisance, de son inefficience, voire de sa « dangerosité » étant donné le mécanisme pollueur-payeur qu'elle entraînera très rapidement. En effet, il y a matière à s'interroger sur le modèle de convention choisi, calqué sur la procédure créée, notamment pour les faits de corruption et de fraude fiscale, par la loi Sapin II en 2016. En reprenant le modèle américain, il s'agit d'ouvrir la possibilité de transaction engagée par le ministère public dans le secteur de l'environnement. Cela permet en réalité de se passer de procès, des droits de la défense et, surtout, d'une véritable reconnaissance de culpabilité. Pourtant, les atteintes à l'environnement pourraient être considérées comme relevant de l'intérêt général, plutôt que de l'intérêt public. Il s'agit désormais d'engager de véritables mesures d'urgence, avec des moyens solides et renforcés, pour lutter contre l'impunité des grands groupes qu'il faut sanctionner en bonne et due forme, plutôt que de préserver en négociant telle amende ou telle réparation de dommage. Ces dommages sont la plupart du temps irrévocables, et non d'ordre financier. Poux réparer une fraude fiscale, on fait payer les fraudeurs ; mais, en matière de pollution, les pollueurs auront beau payer, les dégâts resteront irréversibles. L'actualité en fait malheureusement état chaque nouveau jour qui passe. En outre, ce projet de loi crée des pôles régionaux dans le ressort de chaque cour d'appel. De nouvelles juridictions donc, mais sans moyens supplémentaires, et alors que viennent d'être supprimés les tribunaux d'instance. C'est bien là que le bât blesse. Notre système judiciaire a d'abord besoin de moyens plutôt que de réorganisation, qu'il s'agisse de la Chancellerie ou du ministère de la transition écologique, chargé de la police de l'environnement, dont les moyens en baisse nous laissent craindre une perte d'expertise irrémédiable au sein même des services de l'État. Comment, madame la garde des sceaux, créer les conditions d'une véritable justice environnementale dans ce cadre précaire ? Tout cela résonne d'ailleurs parfaitement avec le projet de loi dit de « simplification de l'action publique », dont l'examen commencera après ces explications de vote. Avec ce texte, présenté trois jours avant la catastrophe de Lubrizol, mais que le Gouvernement n'a pas jugé utile de corriger, le ton est donné. Il s'agit de libérer les entreprises du carcan de contraintes définies par le code de l'environnement, toujours dans la même optique : aller toujours plus vite pour libérer l'économie et la croissance.

je réitère notre opposition à la création de la peine complémentaire d'interdiction d'accès aux transports collectifs. Il ne s'agit, selon nous, que d'une mesure d'affichage tendant une fois encore à instrumentaliser notre droit pénal. La création de nouvelles peines, qu'elles soient complémentaires ou non, est devenue une habitude législative regrettable, toujours dans la même logique : à chaque problème « sociétal » sa réponse pénale, avec un renforcement des peines, sans jamais- je dis -réfléchir à la cohérence d'ensemble de notre système d'échelle des peines, et encore moins aux mesures alternatives de prévention ou de dissuasion. Enfin, vous l'aurez compris, notre groupe ne reviendra pas sur son vote annoncé initialement et s'abstiendra sur ce texte. En effet, les motivations et les compétences actuelles du Parquet européen apparaissent comme assez louables, mais les mesures environnementales fondamentales pour les années à venir sont plus qu'en deçà des attentes de nos concitoyens sur le sujet. Quant aux sujets annexes, sans revenir sur le fond, leur place n'était pas dans le titre III d'un tel texte, dont la cohérence était déjà difficilement lisible dans ses deux volets principaux. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le règlement européen du 12 octobre 2017 a institué un Parquet européen chargé de poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Dans chaque État membre, au moins deux procureurs européens délégués doivent être désignés afin de conduire, sur le plan opérationnel, les enquêtes et de représenter le ministère public devant les juridictions de jugement.

ni les instructions données par le procureur général près la cour d'appel. Il met en oeuvre, en revanche, les orientations arrêtées par le collège du Parquet européen et applique, le cas échéant, ses instructions dans un dossier particulier. Les procureurs européens délégués peuvent exercer les prérogatives reconnues en droit français au procureur de la République, mais aussi prendre des mesures qui relèvent habituellement de la compétence du juge d'instruction, par exemple prononcer une mise en examen. L'organisation d'un Parquet européen hiérarchisé n'est pas compatible avec le statut du juge d'instruction, qui garantit son indépendance et lui interdit de recevoir des instructions. Pourtant,

provisoire. C'est pourquoi le procureur européen délégué pourra conduire les investigations en se situant soit dans le cadre procédural de l'enquête préliminaire ou de l'enquête de flagrance, soit dans le cadre procédural de l'instruction, soit dans ces deux cadres successivement. Cette construction inédite et pragmatique permet de satisfaire aux exigences du droit de l'Union européenne, tout en apportant des modifications d'ampleur limitée au code de procédure pénale puisque ce sont les règles de procédure habituelles, propres à l'enquête ou à l'instruction, qui s'appliqueront. Cette organisation décentralisée n'était toutefois pas celle qui avait été envisagée par la Commission européenne lorsque celle-ci avait présenté, en 2013, sa proposition initiale de règlement portant création du Parquet européen. Ce projet de la Commission était, à l'origine, très intégré un procureur unique aurait disposé d'une compétence exclusive pour mener des enquêtes dans toute l'Union européenne. Ce projet s'est heurté à la ferme opposition de plusieurs États membres. En effet, pour la première fois, 14 chambres parlementaires nationales, dont le Sénat français, ont mis en oeuvre la procédure dite du « carton jaune », estimant que la proposition de la Commission européenne ne respectait pas le principe de subsidiarité. Après quatre années de négociation, nous nous réjouissons qu'un compromis ait été trouvé autour de quelques principes : compétence partagée avec les autorités nationales ; organisation collégiale ; désignation de délégués nationaux chargés de conduire les enquêtes dans chaque État membre. Ce compromis n'a toutefois pas convaincu la totalité des États membres de l'Union européenne, ce qui a justifié de recourir à la procédure dite de coopération renforcée. Y participent 22 États, à l'exclusion de l'Irlande et du Danemark, qui bénéficient d'une clause dite d'« » dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, ainsi que de la Hongrie, de la Pologne et de la Suède, qui ont refusé de s'y joindre. Dans son titre II, ce projet de loi étend les compétences des parquets nationaux spécialisés. Il prévoit la création d'un pôle spécialisé dans le contentieux environnemental dans le ressort de chaque cour d'appel et fixe des règles destinées à régler les conflits de compétences entre juridictions. Ces dispositions ne présentent aucune difficulté. En effet, depuis plusieurs décennies, le législateur a fait le choix de spécialiser des juridictions répressives dans le traitement de certains contentieux, dans le but de traiter avec plus d'efficacité des dossiers techniques ou complexes ou de lutter avec plus de vigueur contre des formes graves de délinquance. À Paris et à Marseille, ont ainsi été créés des pôles compétents en matière sanitaire et environnementale, puis des pôles compétents en matière d'accidents collectifs. En 2004, ont été créées 9 juridictions interrégionales spécialisées, compétentes en matière économique et financière ainsi que pour la criminalité et la délinquance organisées. Plus récemment, des parquets nationaux ont été institués : parquet national financier en 2013 et parquet national antiterroriste en 2019. Le titre II du projet de loi prévoit des dispositifs destinés à régler les conflits de compétences qui peuvent surgir entre ces juridictions spécialisées et les autres juridictions. Il procède également à des aménagements relatifs au parquet national financier et au parquet national antiterroriste et tend à spécialiser certaines juridictions sur le contentieux environnemental afin de mieux réprimer ces infractions. Le groupe Les Indépendants approuve pleinement les dispositions du titre II tout comme celles du titre III, qui comporte notamment des mesures d'adaptation du code de procédure pénale à diverses décisions rendues par le Conseil constitutionnel ou par la Cour de cassation. Je me félicite de ce que, par ses travaux, la commission des lois ait apporté modifications et précisions au projet de loi sans remettre en cause ses équilibres. À cet égard, nous tenons à saluer la qualité des travaux du rapporteur, notre collègue Philippe Bonnecarrère. Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants porte un regard positif sur ce texte et votera ce projet de loi à l'unanimité. Madame Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée.

à monter au plateau pour superviser le déroulement du vote. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter

vous permettez à la fois d'assurer une meilleure efficacité dans la répression des infractions pénales qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union,

le rappelle, si nous avons souhaité transposer aux enjeux environnementaux cette réponse qui existe déjà en matière de fraude, c'est tout simplement parce qu'elle permet d'imposer une amende élevée, qui est extrêmement important. Elle permet également de mettre en place des plans de conformité pour les entreprises. Enfin, elle permet de réparer ou de compenser le préjudice causé.

à incriminer ces comportements par voie réglementaire et, le cas échéant, à confisquer l'aéronef par une peine complémentaire au moment où l'infraction sera commise.

portant sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Lors de ce scrutin, mon collègue Hervé Maurey souhaitait s'abstenir. La parole

Monsieur le président, madame la rapporteure Élisabeth Doineau, madame la rapporteure pour avis Catherine Di Folco, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la perte d'un enfant est une tragédie sans équivalent. Nous avons le devoir d'accompagner le plus et le mieux possible les parents qui sont confrontés à un tel drame. Or, aujourd'hui, à la souffrance des familles s'ajoutent des démarches administratives inextricables, doublées d'inégalités territoriales inacceptables. Comme vous avez eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, madame la rapporteure, l'émotion suscitée par le sort de la proposition de loi du député Guy Bricout a mis en lumière à la fois l'ampleur et la diversité de ces difficultés. Nous devons et voulons y mettre un terme. Mieux, nous devons bâtir un système protecteur et complet. Nous devons bâtir un système dans lequel la douleur de la perte d'un enfant est pleinement reconnue par la société. Un système dans lequel les pouvoirs publics apportent, dans la durée, une réponse à la hauteur des besoins de ces familles endeuillées. Des familles qui, pour reprendre les mots d'une association, « ne sont pas toutes égales dans leurs ressources de résilience C'est précisément ce système, ancré sur la solidarité nationale, qu'il vous est aujourd'hui proposé d'adopter. Il faut souligner que le texte soumis à votre discussion a été considérablement enrichi par rapport à sa version initiale, grâce à un travail de coconstruction inédit, que je salue, et qui s'est matérialisé par le dépôt d'amendements dits « miroir » du Gouvernement. Loin des polémiques, ce qui nous a toutes et tous guidés, ce qui nous guide collectivement, c'est la volonté de créer le plus rapidement possible des droits nouveaux, simples d'accès, pour soulager concrètement les familles, mais aussi amplifier le travail remarquable d'accompagnement mené par les associations au quotidien. Je tiens à saluer cet état d'esprit digne, incarné notamment par la démarche constructive de Mme la rapporteure et confirmée par les commissaires aux affaires sociales. Cette démarche fait écho à la qualité des échanges que nous avons vécus lors des concertations avec les associations et les partenaires sociaux, sociaux, menées conjointement avec mon collègue Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Ces concertations ont été conduites en étroite collaboration avec la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment avec Martin Lévrier, que je salue, mais aussi avec les rapporteurs des deux chambres. Ces concertations s'inscrivent en complémentarité des auditions de la commission, et dans le prolongement des travaux menés en particulier par la sénatrice Catherine Deroche dans le cadre des Assises du deuil que le Palais du Luxembourg a accueillies le 12 avril dernier. Cette mobilisation sans précédent de toutes et tous a permis de dégager rapidement et clairement un plan d'action complet, constitué d'une pluralité d'axes de natures différentes : législative, réglementaire, administrative et conventionnelle. cinq axes forts ont marqué cette proposition de loi de leur empreinte : l'instauration d'un congé de « répit » universel ; le renforcement de la protection contre le licenciement la fin de l'arrêt brutal des prestations familiales et la création d'un parcours administratif facilité ; la création d'une allocation relative aux frais d'obsèques ; et le renforcement de l'accompagnement psychologique. Je développerai les deux premiers, tandis que mon collègue Adrien Taquet présentera les suivants. l'instauration d'un congé de deuil pour tous. La douleur insondable de la perte d'un enfant ne doit pas être différenciée en fonction de statuts : salariés, agents publics- en cela, nous partageons l'intention de la rapporteure pour avis Catherine Di Folco -, indépendants, demandeurs d'emploi. Tous bénéficieront Tous bénéficieront désormais de quinze jours ouvrés de congé de deuil dans le cas du décès d'un enfant jusqu'à l'âge de 25 ans. Au-delà de ce temps, et en fonction de la réaction de chacun, le traumatisme psychologique lié à la perte d'un enfant peut bien sûr pleinement justifier un arrêt de travail pour maladie. Pour éviter des ruptures dans la prise en charge des parents à ce moment, la proposition de loi prévoit désormais que le délai de carence habituellement applicable pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale est supprimé pour le premier arrêt survenant dans les treize semaines suivant le décès. Je m'engage à ce que le délai de carence applicable concernant le versement du complément employeur soit lui aussi supprimé dans les mêmes conditions. Je prendrai un décret en ce sens dès l'entrée en vigueur de la proposition de loi. deuxième axe est le renforcement de la protection des salariés et l'amélioration des conditions de leur retour à l'emploi. Je salue ainsi l'instauration, sur le modèle des dispositions protégeant les mères après un congé de maternité, d'une mesure de protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès de l'enfant. De même, le maintien du mécanisme de don de jours de repos entre salariés, porté par la députée Sereine Mauborgne et voté à l'Assemblée, permettra d'ouvrir une modalité de concrétisation de l'élan de solidarité qui s'exprime entre collègues lors de ces événements tragiques. Si les mesures de précision relevant du champ de la négociation ont été écartées de la proposition de loi, je tiens à souligner à cette tribune les attentes fortes exprimées par les associations vis-à-vis des partenaires sociaux, notamment en matière de retour à l'emploi des parents endeuillés. La mobilisation des partenaires sociaux dans le cadre d'accords d'entreprise ou de branche, constituera un maillon complémentaire à la réponse apportée par l'État, que ce soit en matière de prolongement des aides liées à l'enfant, de création d'une allocation pour les frais d'obsèques ou du renforcement de l'accompagnement psychologique. Je me réjouis de l'adoption, à l'unanimité de la commission, de ces mesures sans précédent, qui constitueront dès leur promulgation des droits concrets pour les familles endeuillées. Nous porterons ces nouveaux droits à l'échelle européenne. Je cède la parole à Adrien Taquet.

Ces dernières semaines nous ont confirmé, chacun dans notre intimité la plus profonde, lors de nos débats et plus encore lors des échanges que nous avons eus avec des parents, que la question du deuil d'un enfant n'exigeait rien d'autre qu'écoute et humilité. Avec la ministre du travail Muriel Pénicaud, en amont de la présentation de ce texte, nous avons réuni les associations à plusieurs reprises, nous avons écouté les familles. Nous voulons les saluer, chacune, et les remercier pour le travail qu'elles effectuent depuis de nombreuses années auprès des parents endeuillés Le Sourire de Lucie, Grandir sans cancer, Naître et vivre, Eva pour la vie, Aidons Marina, l'association Léa, SOS Préma, Apprivoiser l'absence, Mieux traverser le deuil, Empreintes, Jonathan pierres vivantes, Le Point rose ou encore France victimes. D'aucuns auraient pu redouter les échanges avec ces parents, qui ont vécu l'indicible, l'inconcevable, et craindre la douleur, la dureté de ces vies ainsi exposée, cette réalité ainsi bouleversée. Ce fut en réalité tout le contraire tout n'aura été que dignité et placidité, doublées, évidemment, d'une extrême sensibilité à l'égard de ce qui s'est joué, de ce qui a été exprimé. S'il a été une insoutenable dureté lors de ces échanges avec les parents, c'est bien celle qui a consisté à toucher du doigt l'incapacité des pouvoirs publics jusqu'à présent

d'imaginer un accompagnement qui soit, tout simplement, digne, c'est-à-dire à la hauteur de la dignité des parents eux-mêmes. Il était important, tout d'abord, d'allonger la période de répit dont peuvent disposer les parents après le décès de leur enfant. Ainsi, comme la commission en a décidé au travers de l'adoption d'un amendement de Mme la rapporteure, cette période sera désormais portée à quinze jours : sept pris en charge par l'employeur- Muriel Pénicaud l'a rappelé -et huit pris en charge par la solidarité nationale, la branche famille de la sécurité sociale.

ou non-salariés agricoles. Quant aux demandeurs d'emploi, ils seront, pendant cette période, dispensés de recherche mais continueront de percevoir leurs allocations. Chacun de nos enfants est différent ; chaque histoire que nous avons nouée avec eux est différente ; chaque douleur est différente ; toutefois, tous les parents endeuillés doivent pouvoir disposer des mêmes garanties de répit, afin de commencer, tout doucement, à faire face

sur le plan administratif, financier et psychologique, mais aussi dans le regard que ceux qui les entourent, que la société portent sur elles. il fallait également que ce congé de répit s'inscrive dans un cadre élargi prévoyant le prolongement, pendant trois mois, du versement des prestations : les allocations familiales, le complément familial, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

en compte dans le calcul du RSA et de la prime d'activité. Ce texte permettra également aux parents qui ne peuvent pas reprendre le travail après un deuil de ne pas subir le délai de carence attaché au congé maladie ; Mme la ministre du travail l'a indiqué. Le choc induit par le deuil ne doit pas effacer les problèmes financiers auxquels se trouvent confrontées certaines familles pour prendre en charge les frais de funérailles de leur enfant. Des témoignages poignants nous ont permis de réaliser ce que c'était parfois le cas et que seul le soutien des associations permettait de sortir de ces difficultés. ce n'est pas le rôle de ces associations ; il revient, là aussi, à la solidarité nationale d'être aux côtés des parents endeuillés ; ainsi, une prestation forfaitaire et universelle sera versée en cas de décès de l'enfant afin de couvrir, notamment, les frais d'obsèques. Le versement de cette prestation sera automatique pour les allocataires des caisses et sera très facile d'accès- sur simple demande -pour les autres. Le montant de cette prestation sera défini dans un décret que nous soumettrons à la concertation. Les caisses d'allocations familiales (CAF) sont d'ores et déjà pleinement mobilisées pour accompagner les parents, dans le cadre du parcours deuil qu'elles ont mis en place ; elles le resteront évidemment et elles veilleront à alléger autant que possible les démarches administratives qui doivent être accomplies en un tel cas. Je m'y engage cas. Je m'y engage personnellement et je sais pouvoir compter sur Vincent Mazauric, le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales, pour mettre tout en oeuvre à cet effet, en s'appuyant tant sur le personnel des caisses et les travailleurs sociaux que sur le tissu associatif, dont nous connaissons le rôle indispensable. Enfin, nous devons également assurer un accompagnement psychologique aux familles touchées par le deuil d'un des leurs. Le deuil est le drame d'une vie ; il touche non seulement les parents mais aussi l'ensemble de la famille, notamment les frères et les soeurs. Chaque membre de la famille doit pouvoir trouver un soutien approprié. Ainsi, un accompagnement psychologique de plein droit sera proposé, afin que les familles qui le souhaitent puissent bénéficier de l'aide et de l'écoute de professionnels, en fonction de leurs besoins. Mesdames, messieurs les sénateurs, grâce à ce texte, grâce au travail sans relâche des associations et grâce aux nouvelles propositions des députés et des sénateurs, nous avons aujourd'hui la possibilité de faire de la France un pays en pointe, dont pourraient s'inspirer certains de nos voisins européens, à commencer par la Belgique, qui débat de ce sujet en ce moment

accepter que l'enfant que l'on a aimé ne reviendra plus et réapprendre à vivre ». Je tiens à remercier sincèrement, une nouvelle fois, les associations de leurs actions primordiales en faveur de tous les parents endeuillés, de leur temps et de leurs propositions, qui inspirent le texte débattu aujourd'hui. Je veux aussi remercier les parlementaires tous ensemble, essayons d'apporter le soutien de la Nation à ces familles. Au-delà, tâchons de sortir ce sujet de l'ombre, car c'est aussi de cela qu'il s'agit, mesdames, messieurs les sénateurs ; par nos échanges, nous contribuons à faire tomber un tabou, celui de la mort d'un enfant ; c'est ce que les familles appelaient de leurs voeux depuis longtemps. Par nos échanges, nous faisons sortir de l'ombre non seulement la question de la mort d'un enfant, mais encore des milliers de familles qui, désormais, peuvent espérer être mieux comprises par ceux qui les entourent. nous devons garder toujours en tête quelque chose que nous n'avions peut-être pas perçu, que la société tout entière n'a probablement pas compris : quand on est parent, on l'est pour la vie, par-delà la mort. La parole

Rien n'est pire pour des parents que de perdre un enfant. La proposition de loi de notre collègue député Guy Bricout, qui est présent faisait écho à l'histoire de Pascaline, une maman à jamais marquée par un tel drame. Notre collègue pensait- on peut le comprendre -que sa proposition de loi tendant à porter de cinq à douze jours le congé prévu par le code du travail en cas de décès d'un enfant mineur ferait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été le cas, ce qui a provoqué une indignation légitime des parents concernés et de l'opinion en général.

; notons une célérité inhabituelle pour un texte qui n'émane pas des rangs de la majorité ! Néanmoins, réjouissons-nous, ce sujet méritait une ambition commune, transpartisane et unanime. Permettez-moi de le souligner : cet épisode constitue une nouvelle illustration de l'importance du bicamérisme et de l'utilité du Sénat. La commission des affaires sociales de la Haute Assemblée a ainsi abouti, avec l'accord du Gouvernement, à un texte permettant non seulement d'instituer de nouveaux droits en cas de décès d'un enfant, mais encore d'améliorer l'accompagnement des familles endeuillées. Je l'ai indiqué, le texte initial de notre collègue député Guy Bricout consistait en une proposition simple ; contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, celle-ci n'était pas mal ficelée, était limitée par l'article 40 de la Constitution. Le texte transmis par l'Assemblée nationale au terme de ses travaux comportait deux articles. Plutôt que d'allonger la durée du congé pour décès d'un enfant,

Une telle disposition n'avait qu'une portée indicative, puisqu'un tel accord collectif peut actuellement être conclu sans qu'une habilitation législative soit nécessaire. En outre, cette proposition posait des difficultés juridiques non négligeables, par exemple dans les entreprises dans lesquelles les congés annuels sont imposés. J'ajoute que cette disposition aurait été sans effet pour les salariés perdant un enfant et ayant déjà pris tous leurs congés annuels.

Si l'intention était louable, un dispositif de don de jours peut difficilement être mobilisé immédiatement après le décès d'un enfant et il exige une démarche, au succès incertain, de la part du salarié concerné. Surtout, un tel dispositif ne peut bénéficier de la même manière à tous les salariés, selon la taille de leur entreprise. Le texte qu'il nous était donné d'examiner ne répondait donc que très marginalement aux besoins des familles et, malgré un dispositif juridique plus complexe, il était en deçà de l'ambition initiale de la proposition de loi. Je dois ici faire justice au Gouvernement en reconnaissant qu'il a bien pris conscience de cette insuffisance et que la ministre du travail comme le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance ont souhaité contribuer utilement au travail de la commission des affaires sociales, afin de sortir par le haut de la polémique née à l'Assemblée nationale. Le texte issu des travaux de la commission, complété par ceux de la commission des lois, dont je salue le rapporteur pour avis, Catherine Di Folco, comprend désormais neuf articles, issus d'initiatives de sénateurs de différents groupes, en coopération avec le Gouvernement, lequel a pu lever l'irrecevabilité financière. de l'article 1, la commission est revenue à l'esprit initial du texte, tout en allant plus loin. Tout travailleur, salarié ou indépendant, qui perd un enfant âgé de moins de 25 ans aurait ainsi droit à quinze jours de congé. Pour les salariés, les sept premiers jours ouvrés- les cinq jours actuellement prévus par le code du travail augmentés de deux -seraient rémunérés par l'employeur les huit jours suivants pourraient être pris dans l'année suivant le décès, de manière fractionnée, et ils feraient l'objet d'une indemnité journalière de la sécurité sociale, complétée par l'employeur à hauteur du salaire.

Ce droit serait ouvert pour le décès d'un enfant du travailleur concerné jusqu'à 25 ans. Certains auraient préféré inclure les enfants à charge sans lien de filiation, afin de tenir compte des familles recomposées, mais le Gouvernement en a arbitré différemment. L'article 1 , issu d'un amendement de la commission des lois, instaure un dispositif équivalent pour les fonctionnaires ; je laisserai le rapporteur pour À l'article 2, nous avons précisé le dispositif de don de jours de congé, afin notamment de définir la période pendant laquelle il peut être mobilisé : une année. Un amendement de la commission des lois a prévu son extension aux fonctionnaires. L'article 3 est issu de travaux menés par notre collègue Catherine Deroche. Il propose de maintenir plusieurs prestations familiales pendant une période déterminée par décret. Il est évident que les dépenses à la charge des parents ne se réduisent pas brusquement avec le décès d'un enfant. Ce maintien, pendant une période qui devrait être de trois mois, doit permettre de ne pas ajouter des difficultés financières à la douleur considérable des parents. L'article 4, proposé également par Catherine Deroche, crée une allocation forfaitaire versée automatiquement et destinée à aider au paiement des frais d'obsèques. Le montant de cette allocation, fixé par décret, sera modulé en fonction du revenu du foyer et pourra être complété par les caisses au titre de leur action sociale. Je laisserai le Gouvernement préciser son intention, les associations étant un peu déçues. L'article 5, issu d'un amendement de notre collègue Martin Lévrier, propose une mesure similaire pour ce qui concerne le revenu de solidarité active et la prime d'activité. L'article 6, que nous avons également adopté sur proposition de Martin Lévrier, prévoit une expérimentation portant sur la prise en charge de la souffrance psychique de la famille d'un enfant décédé. Il me semble que cette mesure est de nature à répondre à la demande forte d'accompagnement médico-social et psychologique formulée par les associations de parents. De mon côté, j'ai souhaité compléter la proposition de loi afin de tenir compte des demandes exprimées par les associations que j'ai rencontrées. L'article 7 introduit ainsi une protection contre le licenciement des salariés ayant perdu un enfant, pendant une durée de treize semaines, à l'instar de ce dont bénéficient les jeunes mères. Les organisations patronales ne sont pas opposées à cette mesure. Enfin, l'article 8 supprime le délai de carence pour le premier arrêt maladie qui suit le décès d'un enfant, et ce pour la même durée de treize semaines. Le choc représenté par la perte d'un enfant peut rendre la reprise du travail impossible, même après une période de congé. De nombreux salariés sont alors mis en arrêt de travail par leur médecin. Imposer des jours de carence avant le versement d'indemnités journalières en pareil cas paraît inhumain.

Les associations que nous avons, les uns et les autres, rencontrées avancent la nécessité de mettre en place un réel parcours de deuil pour accompagner les familles. Ce parcours doit être personnalisé, car chacun ne vit pas la douleur de la même manière.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des lois a souhaité se saisir pour avis de la proposition de loi déposée par notre collègue député Guy Bricout, afin de permettre aux agents publics de bénéficier des mêmes garanties que celles qui sont prévues pour les salariés de droit privé, dans une situation particulièrement douloureuse. Quelles sont les différences entre le secteur public et le secteur privé ? Lorsqu'ils perdent un membre de leur famille, les agents publics peuvent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence (ASA). La durée de celles-ci varie toutefois d'une fonction publiques hospitalière et territoriale, la durée des ASA est laissée à la libre appréciation des employeurs ; chaque collectivité territoriale délibère sur sa propre doctrine.

ces autorisations constituent non pas un droit, mais une simple « mesure de bienveillance » de la part de l'administration, que les chefs de service peuvent accorder à titre facultatif, contrairement à ce qui Cette durée de trois jours est donc inférieure au congé de deuil dans le secteur privé. Dans le secteur public, les autorisations spéciales d'absence sont assimilées à un temps de travail effectif mais ne produisent aucun droit à congé payé, contrairement à ce qu'il se passe dans le secteur privé ; en outre, les agents peuvent perdre certaines de leurs primes. La proposition de loi de notre collègue Bricout a été malmenée à l'Assemblée nationale. Le texte issu de la première lecture constitue une occasion manquée à un double titre : avec l'accord du Gouvernement, les députés ont supprimé l'allongement du congé de deuil dans le secteur privé et ils ne se sont pas préoccupés des 5,33 millions d'agents publics, qui représentent pourtant 21 % de la population active. Nous souhaitons donc, à la faveur de l'examen du texte par la Haute Assemblée, corriger ces deux lacunes afin de mieux accompagner les parents endeuillés. Du reste, les employeurs publics que j'ai auditionnés semblent tout à fait favorables à cette manifestation de solidarité. La commission des lois a adopté deux amendements visant à offrir les mêmes garanties aux agents publics- fonctionnaires ou contractuels -qu'aux salariés de droit privé. Le premier amendement avait pour objet de recourir aux ASA sans qu'il soit besoin de créer de nouveaux congés. plus simple du point de vue juridique, permet d'appliquer la mesure à l'ensemble des catégories d'agents publics, y compris lorsqu'ils sont contractuels. Il était prévu une première autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrés, quel que soit l'âge de l'enfant, au moment du décès, sans possibilité de fractionnement, et une seconde, de dix jours ouvrables, lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ou à charge. Cette seconde ASA pouvait être fractionnée, dans un délai de six mois à compter du décès, les jours non consommés ne pouvant être reportés ni figurer dans un compte épargne-temps. Ces autorisations spéciales d'absence étaient accordées de droit et étaient assimilées à un temps de travail effectif, les agents conservant leur traitement indiciaire ainsi que leurs droits à formation et à la retraite. Par cohérence avec le secteur privé, elles entraient également en compte pour le calcul des congés payés.

Le Gouvernement a prévu de prendre en charge une partie des autorisations d'absence, dans des conditions définies par décret. Pour que les choses soient plus claires, pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'État, préciser le dispositif envisagé pour la fonction publique

de ces derniers. Il est conséquent pour les familles recomposées, de plus en plus nombreuses, car il couvre les enfants du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin. Certains de mes amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. Toutefois, a finalement déposé des amendements visant à inclure les enfants à charge dans l'ensemble des dispositifs ; je me réjouis que mes arguments aient été entendus et je vous remercie, madame la ministre, monsieur le secrétaire Le second amendement de la commission des lois visait à autoriser les agents civils et militaires à donner des jours de repos ; il a été intégré au texte de la commission, je vous en remercie, madame la rapporteure. Néanmoins, il serait utile de simplifier les procédures, afin d'encourager les agents publics à donner des jours de repos. Certaines règles semblent, en effet, superfétatoires, comme la nécessité d'obtenir l'accord de son chef de service. Une simple obligation d'information pourrait suffire, sans que cela remette en cause le bon fonctionnement du service. C'est ce que je vous proposerai au cours de l'examen du texte. La parole est à M.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire il est des moments de grâce que l'on ne saurait bouder, de grands moments où l'humanité et l'empathie l'emportent sur toute autre considération, au-delà des différences de sensibilité. Dès qu'a été connu le rejet de la proposition de Guy Bricout, nos concitoyens, quel que soit leur statut social ou professionnel, quelle que soit leur appartenance politique ou syndicale, ont exprimé leur incompréhension et leur générosité, une générosité qui se manifeste toujours dans les grands moments et dont il ne faut jamais désespérer. Ils se sont exprimés par milliers pour dire, avec leur coeur, que la Nation doit apporter à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui souffrent de la plus tragique des séparations, sa sympathie et son soutien, par des actes qui soulagent, qui accompagnent, et qu'elle doit- avec toute la délicatesse nécessaire -prendre en charge tout ce qui, en de tels moments, complique douloureusement le quotidien.

n'était pas, tant s'en faut, des plus simples. Pas simple de donner une suite décente et globale à la proposition de loi transmise sous une forme si édulcorée par l'Assemblée nationale et d'élaborer un texte à la hauteur des attentes Pas simple de formuler des propositions issues d'une appréciation globale des situations de détresse, d'élaborer des propositions embrassant la totalité des besoins exprimés ou implicites, tout en évitant deux écueils, celui de la surenchère- particulièrement inopportune et indigne -et celui des bonnes intentions parfois toxiques, qui peuvent être intrusives quand elles viennent bouleverser plus encore une famille désemparée

Ne restait, pour les salariés désemparés, que le droit opposable à l'employeur, de prélever une partie des congés ou des RTT. Ainsi, faute de disposer du pouvoir de créer des recettes, le Sénat risquait de voir repousser toutes ses initiatives. C'est

C'est dans ce contexte, assurément surréaliste, qu'ont pu sortir du néant des moyens cohérents avec nos ambitions et plus humains, lesquels recueillent notre adhésion pleine et entière. Engagés dans cette volonté commune d'apporter réconfort, soulagement et accompagnement,

Le congé serait porté à douze jours ouvrés sur trois semaines, sécables en fonction du souhait des salariés. La prise en charge des frais d'obsèques serait assurée selon un forfait de portée nationale ; ce forfait doit comprendre, selon nous, frais engagés pour le recours éventuel à des aides à domicile, si la famille en éprouve le besoin. C'est aussi un geste tout en délicatesse et réaliste que cette disposition de versement prolongé, au-delà du décès, des prestations familiales, éviter que la rupture soit aggravée par une violence supplémentaire et que l'administration soit conduite à envoyer des courriers intempestifs et brutaux sitôt le décès

Mon intention n'est évidemment pas de détailler les propositions de la commission ; cela a été excellemment fait et le document qui nous a été remis est suffisamment explicite et détaillé. Hélas, la prise en charge de l'accompagnement psychologique a été oubliée par le Gouvernement, malgré ses belles déclarations ! Oubli ou volonté malvenue de réaliser quelques économies ? En tout cas, un amendement judicieux est venu contourner la difficulté du financement par le biais du recours à une expérimentation. Ainsi, puisqu'il faut en passer par un artifice pour combler une lacune, acceptons-en la rédaction. Sans doute la loi ne peut-elle tout dire, notamment sur l'environnement humain au travail, sur l'intérêt qu'il y a ou non à changer de poste ou à imaginer une reprise modulée. Les accords d'entreprise ou de branche devraient, nous l'espérons, y pourvoir ;

pour l'équilibre de nos institutions que le Gouvernement veuille s'approprier le monopole des réformes quitte à s'opposer aux propositions du Parlement, au détriment de ceux à qui ces réformes devraient profiter.

Or- cela pourrait être risible -c'est l'un des seuls cas où le système actuel est préservé et où, justement, le système à points ne s'applique pas. L'aide aux aidants de notre collègue Jocelyne Guidez avait été votée à l'unanimité par notre assemblée et repoussée au motif que le Gouvernement allait proposer mieux. Il l'a proposée, mais avec une importante économie de moyens Notre pays est au bord de l'explosion. Il n'en peut plus des déclarations grandiloquentes aux effets dérisoires. Il n'en peut plus de l'accroissement des inégalités. Il n'en peut plus de ce mépris affiché à l'égard du Parlement, auquel on présente un projet de réforme du système de retraites plein de trous, sans en révéler le coût monstrueux et les profondes injustices potentielles, et dont on interrompt les débats par un 49-3 brutal, alors qu'il suffisait de se donner le temps. Quel rapport ? Hors sujet ! L'arrêt des débats intervient juste- est-ce un hasard ?

Ces changements de pied, ces blocages, ces prétextes pour ne pas débattre au fond de projets mal préparés, ce sentiment donné aux Françaises et aux Français que le pouvoir est concentré en une seule paire de mains contribuent à discréditer les institutions chargées de les représenter. Le Sénat, qui débat et débattra avec sérieux et sens de la mesure, démontrera de nouveau combien il est un outil essentiel de la démocratie. N'étant inféodé à personne, il a toujours affiché sa liberté de penser, tout au long de son histoire. Le général de Gaulle lui-même, qui, pourtant, lui avait donné ses prérogatives et ses lettres de noblesse, a fait l'amère expérience d'une volonté d'indépendance qui ne se négocie pas

évidente : « Ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. »

Est-il nécessaire de rappeler que chaque année, en France, près de 4 500 enfants décèdent avant d'avoir atteint l'âge de la majorité ? Par ailleurs, en 2017, selon les données de l'Insee, ce sont près de 6 500 enfants et jeunes de moins de 25 ans qui sont décédés, dont 2 700 âgés de moins de 1 an et 2 400 âgés de 15 à 24 ans. La douleur liée à la perte d'un être cher est incommensurable. Si l'on y ajoute les les démarches administratives, l'organisation des funérailles, le deuil, les parents concernés ne sont généralement pas en mesure de reprendre leur travail à l'issue des cinq jours prévus par la loi. Mes chers collègues, Actuellement, en application de l'article L. 3142-4 du code du travail, les salariés dont l'enfant décède disposent uniquement d'un congé de cinq jours, pris en charge par l'employeur. Il est évident que, sur le plan émotionnel et d'un point de vue pratique, une telle durée est très insuffisante. En effet, En effet, cette période de congé permet tout d'abord aux parents endeuillés d'accomplir les démarches qui s'imposent après le décès, telles que l'organisation des obsèques ou encore la mise à jour du livret de famille. Même si l'on ne peut évaluer la durée du congé qui serait nécessaire pour faire face à la perte d'un enfant, il est indispensable que les parents s'accordent un temps de répit avant de reprendre leurs activités professionnelles. C'est en partant de ce constat que notre collègue député Guy Bricout, que je salue, a proposé de porter la durée de ce congé de cinq à douze jours consécutifs. Il estime, et nous le rejoignons, que le congé de cinq jours prévu en cas de décès d'un enfant est insuffisant pour permettre aux parents « de surmonter ce terrible moment, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue des funérailles et,, pour régler toutes les formalités pratiques et administratives Les besoins des familles endeuillées ne sont pas les mêmes selon les situations, sociale ou financière, dans lesquelles elles se trouvent. Je tiens aussi à souligner que, même si de nombreux salariés bénéficient de la bienveillance de leur employeur et de leurs collègues, d'autres n'ont d'autre choix que de prendre des jours de congé décomptés de leur temps de congé annuel ou de demander un arrêt maladie à leur médecin. Il est quelque peu immoral qu'un parent endeuillé ait à recourir à pareille alternative afin de récupérer émotionnellement avant la reprise de son travail. vous comprendrez pourquoi nous déplorons l'adoption, par l'Assemblée nationale, le 30 janvier dernier, d'un texte ne répondant pas convenablement aux ambitions initiales de son auteur. Cette nouvelle version a suscité une grande émotion, tout à fait compréhensible, des parents concernés, une indignation de la classe politique et de l'opinion publique et une réaction du Gouvernement, qui a souhaité que le texte soit amélioré, après que le Président de la République lui a demandé de « faire preuve d'humanité ». L'humanité est un marqueur du Sénat. Oui, mes chers collègues, nous devons en faire preuve. C'est pourquoi le groupe RDSE se félicite de ce que la commission des affaires sociales ait adopté, à l'unanimité, un texte qui améliore « les droits d'absence des salariés à la suite du décès d'un enfant,

et opérant. Il est vrai, cependant, que le coût du dispositif proposé reposait entièrement sur les entreprises, comme l'a relevé Mme la ministre du travail. Par ailleurs, il n'est pas très judicieux de supprimer l'instauration d'un congé de deuil de douze jours pour la la remplacer par la possibilité ouverte aux partenaires sociaux de conclure une convention ou un accord ouvrant au salarié le droit de prendre les congés payés et les jours de RTT qu'il a acquis dans la foulée du congé pour décès d'un enfant. En conditionnant à un accord d'entreprise ou de branche le droit de prendre des congés payés ou des jours de RTT après un congé pour décès d'un enfant, la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est bien en deçà de la rédaction du texte issu des travaux de sa commission, qui garantissait garantissait à tous les salariés au moins le droit de prendre des jours de congé à la suite d'un congé de deuil. Face à la polémique, madame la ministre, vous avez reconnu une « erreur collective » et, monsieur le secrétaire d'État, vous avez annoncé le lancement d'une concertation pour améliorer les mesures de soutien aux parents endeuillés par la mort d'un enfant. La commission des affaires sociales du Sénat a incontestablement fait preuve d'humanité sur plusieurs points. Tout d'abord, concernant l'article 1, la commission, sur proposition de notre rapporteure Élisabeth Doineau et du Gouvernement, a porté de cinq à sept jours la durée du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Elle a, par ailleurs, créé un « congé de répit » de huit jours, pendant lesquels le salarié bénéficierait d'une indemnité journalière de la sécurité sociale. Pour les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et les demandeurs d'emploi, qui ne bénéficient pas de l'autorisation d'absence financée par l'employeur, la durée du congé est portée à quinze jours et peut être fractionnée, de manière à atteindre la même durée globale que celle qui est accordée aux salariés. Je salue aussi l'adoption par la commission d'un article additionnel après l'article 1, qui prévoit d'étendre les dispositions de la proposition de loi aux fonctionnaires et aux agents contractuels. S'agissant de l'article 2, la commission a estimé que le dispositif de don de jours de repos n'était pas facilement mobilisable immédiatement après le décès d'un enfant. Aussi, sur proposition des deux rapporteurs, elle a défini une période d'un an pendant laquelle ce mécanisme pourrait être utilisé au profit d'un parent endeuillé. Par souci d'harmonisation avec l'article 1, la limite d'âge des enfants concernés a été portée de 20 à 25 ans et le dispositif a été étendu aux agents publics. Nous nous félicitons de ce que notre commission ait introduit plusieurs articles pour améliorer les droits sociaux des familles endeuillées. Même si de nombreuses situations trouvent une solution dans le cadre de la relation du salarié avec son employeur, il est souhaitable de garantir un temps de répit correct pour tous les salariés et de l'harmoniser, dans la mesure du possible, pour l'ensemble des actifs. Nous devons réfléchir à la manière dont les familles endeuillées devront être mieux accompagnées, car les circonstances des décès ne sont pas les mêmes selon les situations et nous réagissons forcément tous de manière différente. Cela doit être pris en compte dans le texte qui nous sera soumis. Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE sera favorable à cette proposition de loi, avec les aménagements proposés.

Permettez-moi de citer Christian Bobin : « Pour être dans une solitude absolue, il faut aimer d'un amour absolu. » C'est bien cette tragédie de la solitude absolue ont à affronter. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet hémicycle pour examiner la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d'un enfant. Déposé par notre collègue député Guy Bricout et le groupe UDI, Agir et Indépendants, ce texte comportait initialement un article unique, lequel visait à allonger le nombre de jours de congé légalement octroyés lors de la survenance d'un décès d'un enfant mineur, le faisant passer de cinq à douze jours successifs. Chacun connaît le contexte particulier dans lequel nous avons été saisis de ce texte. Avant d'aller plus loin, je tenais avant tout à exprimer ma compréhension de l'émoi suscité par les débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier Il n'existe pas de bonnes réponses à l'indicible. La législation ne fait pas exception. Qui serions-nous pour nous indigner des maladresses qu'il a pu y avoir sur les bancs de l'Assemblée nationale ? Qui serions-nous pour imaginer que qui que ce soit puisse être insensible à la nouvelle de la mort d'un enfant ? enfant ? Au reste, ces maladresses ont permis de mettre en lumière les difficultés et le besoin d'accompagnement de la part des pouvoirs publics, en complément de l'action du tissu associatif, qui est très présent sur ces questions et dont je salue le travail. Ce sont les associations qui nous ont montré combien les démarches administratives pouvaient ajouter de la souffrance à la souffrance et à quel point l'absence des pouvoirs publics à cette période était flagrante.

Ces concertations ont permis de dégager six pistes de réflexion : un répit de deuil de quinze jours ouvrés, une aide financière aux obsèques de l'enfant, un parcours administratif facilité, un accompagnement psychologique de plein droit, une protection contre le licenciement et une adaptation des conditions de travail, une sensibilisation sociétale au deuil. Ce travail a été remis à Mme la rapporteure. Il est venu en complément des auditions que celle-ci a effectuées dans le cadre de sa mission. J'en profite pour souligner le travail remarquable qu'elle a réalisé, en parfaite intelligence et dans un consensus transpartisan. Tout en louant ce travail, la commission des affaires sociales a adopté un certain nombre d'amendements. Il me paraît important d'en rappeler les points saillants : l'allongement de cinq à quinze jours du congé de deuil pour le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans-

l'application de ce dispositif de manière universelle, aussi bien aux fonctionnaires qu'aux actifs non salariés ; une aide financière universelle versée par l'État, à laquelle s'ajoutera une aide modulable versée par les CAF afin de participer aux coûts des obsèques le maintien des prestations familiales jusqu'à trois mois après le décès ; l'automaticité du maintien de la prise en compte de l'enfant décédé dans le calcul du RSA ; l'expérimentation permettant la prise en charge par l'assurance maladie d'un accompagnement psychologique lorsque les parents ou les frères et soeurs en font la demande la protection contre le licenciement jusqu'à treize semaines suivant le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, en plein accord avec les organisations patronales. La présente proposition de loi vise à permettre aux parents qui vivent un tel drame d'entamer un travail de deuil sans subir de contraintes administratives disproportionnées et tend, dans la mesure du possible, à alléger le poids financier lié au décès. Pour autant, il me paraît important d'insister sur la nécessité d'étudier le retour au travail pour les parents qui ont été confrontés à cette perte. n'a pas été retenue par la commission, était d'inviter les partenaires sociaux à réfléchir ensemble sur ce point. Malgré un début d'examen chaotique, ce texte démontre que, sur un sujet aussi sensible,

Pour être dans une solitude absolue, il faut aimer d'un amour absolu. » Souhaitons que cette proposition de loi mette en évidence combien la Nation se doit d'accompagner celles et ceux qui subissent cette indicible souffrance.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est peu de dire que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui aura fait couler beaucoup d'encre et suscité un émoi très important, en raison de l'attitude peu glorieuse- les mots sont faibles -du Gouvernement et des députés de La République En Marche lors de son examen à l'Assemblée nationale. Ce texte, originellement destiné à allonger les droits d'absence des salariés après le décès d'un enfant, y a été vidé de son contenu avant d'être renvoyé à notre commission des affaires sociales.

Désormais, nous pouvons dire que nous avons un texte à la hauteur des attentes de la société et des parents qui éprouvent directement ou indirectement cette situation tragique qu'est la perte d'un enfant. Nous y sommes, pour notre part, d'autant plus sensibles que nous défendons depuis très longtemps l'instauration d'un congé de deuil comme une exigence humanitaire parmi les plus élémentaires. En effet, c'est le ministre communiste Anicet Le Pors, dans sa loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui a, pour la première fois, créé, dans la fonction publique, une autorisation spéciale d'absence de deux jours en cas de décès. En 2016, lors de l'examen de la loi Travail au Sénat, notre groupe avait fait adopter un amendement tendant à allonger de deux à trois jours le congé en cas de décès du conjoint ou d'un membre de la famille.

Désormais, les salariés, les travailleuses et les travailleurs indépendants et les agents de la fonction publique bénéficieront d'un congé en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, financé par les entreprises. Nous espérons que les collectivités territoriales et les entreprises qui ont des accords collectifs plus favorables joueront le jeu, en maintenant leurs dispositifs complémentaires. Une nouveauté est proposée avec la création d'un congé de répit de huit jours, fractionnable sur l'année pour permettre aux familles de faire leur deuil. Ces huit jours seront pris en charge par la sécurité sociale sous la forme d'une indemnité journalière. La création de ce congé de répit est positive, mais nous alertons sur les risques que pourrait entraîner cette disposition si le Gouvernement continue de ne pas compenser intégralement les exonérations de cotisations sociales à la sécurité sociale. Nous souhaiterions avoir des garanties que le Gouvernement, si disposé aujourd'hui à faire financer ce dispositif de solidarité par la sécurité sociale, donc par les cotisations des salariés et des employeurs, compensera intégralement ces exonérations. Sinon, cette Sinon, cette mesure serait non seulement de l'affichage, mais une coquille vide. Nous saluons, enfin, les autres mesures complémentaires du texte, qui vont dans le sens du progrès, qu'il s'agisse de la protection des salariés contre le licenciement après le décès d'un enfant, de la suppression des jours de carence, que nous souhaitons généraliser par ailleurs, de la création d'une prestation forfaitaire de 1 500 euros pour les frais funéraires ou encore du maintien des prestations familiales trois mois après la disparition de l'enfant. je ne peux terminer mon intervention sans revenir sur ce qui a été présenté comme une « erreur » du Gouvernement lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale. Peut-on vraiment parler d'« erreur » Nous pensons, au contraire, que, ce qui s'est passé, loin d'être une « erreur », est un « révélateur » de la véritable identité de La République En Marche, pour qui la finance comptera toujours plus que l'humain.

déjà, notre ministre voulait priver les personnes âgées d'exonérations de cotisations pour l'emploi d'une aide à domicile ? Ce n'est donc pas un « dérapage » ou une « erreur ». Il s'agit bien d'une ligne de conduite pleinement assumée,

part, nous prenons nos responsabilités, en considérant que, si aucun délai ne sera à la hauteur de ce que les parents vivent, cette proposition de loi améliore l'accompagnement des familles dans ces moments tragiques. Pour cette raison, et parce que c'est la seule qui importe, le groupe CRCE votera en faveur de ce texte. Madame Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis heureux de saluer la présence, dans nos tribunes, des auditrices et des auditeurs de la cinquième promotion de l'Institut du Sénat. l'initiative de notre ancien collègue Jean Léonce Dupont, le bureau du Sénat avait décidé, en 2015, de mettre en oeuvre ce programme de formation, en vue de mieux faire connaître les modalités de fonctionnement et les enjeux de notre démocratie parlementaire à des personnalités d'horizons géographiques et professionnels très divers. auditeurs de cette cinquième promotion, venant de plus de quinze départements et collectivités d'outre-mer différents, représentent en effet toutes les sphères d'activité professionnelle : publique, économique, sociale, associative, syndicale ou encore universitaire. Tout au long de leurs travaux, qui ont commencé ce matin et s'achèveront à la fin du mois de juin, ils rencontreront plusieurs de nos collègues sénateurs et des fonctionnaires du Sénat. En votre nom à tous, je leur souhaite une excellente session au Sénat et je suis certain que, à l'issue de ces trois mois, ils pourront être les témoins privilégiés de la place essentielle de notre institution au sein de la V République et de la qualité du travail parlementaire.

y a-t-il plus douloureuse épreuve, dans une famille, que la perte d'un enfant ? Celle-ci est un terrible choc. Puis vient le temps des nombreuses démarches, du deuil et de la reconstruction. Améliorer l'accompagnement des parents qui y sont confrontés est l'objet de la proposition de loi déposée par le député Guy Bricout, dont nous ne pouvons que saluer l'initiative. Ce texte vise à porter à douze jours le congé d'un parent salarié venant de perdre son enfant. Ce congé très spécifique était, à l'origine, de deux jours seulement, avant l'adoption de la loi du 8 août 2016, qui a étendu ce droit à cinq jours, sans condition d'ancienneté et sans réduction de rémunération. Avoir plus de temps pour gérer la dimension pratique du décès d'un enfant, se préparer plus paisiblement n'est pas un luxe. Or certains parents endeuillés ne peuvent pas se permettre de prendre plus que ce que la loi accorde. Chez nos voisins, la Suède propose un congé de dix jours. Le Royaume-Uni offre deux semaines. Bien sûr, chaque personne est libre de prendre ces congés ; cela n'a rien d'une obligation. D'ailleurs, certains parents préféreront reprendre le travail rapidement, pour mieux affronter l'épreuve. Il me semble que la meilleure réponse est celle qui saura s'adapter aux besoins de chacun. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a souhaité remplacer l'article unique de la proposition de loi par l'ouverture d'un droit au congé au bénéfice du salarié, dans la limite des jours qui lui sont accordés. Cette position n'est pas en phase avec la réalité. De la même façon, il ne paraît pas opportun de remplacer ces sept jours de congé supplémentaires par un dispositif de don de jours de congé de la part d'un autre salarié de l'entreprise. Il est normal que la solidarité s'exerce en priorité de la part de l'entreprise vis-à-vis de son salarié, avant de s'exercer entre salariés. Aussi, le don de jours de repos est un dispositif intéressant, mais qui ne peut être que complémentaire au droit au repos des parents. Les deux commissions sénatoriales ont amélioré le texte afin de faciliter au mieux la vie des parents endeuillés et d'améliorer leurs droits sociaux. La commission des affaires sociales va plus loin que le texte initial, en portant le droit au congé à quinze jours pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans. La prise en charge des sept premiers jours de congé sera assurée par l'entreprise. Par ailleurs, la commission a adopté un amendement déposé par le Gouvernement, tendant à créer un nouveau congé de répit, d'une durée de huit jours, fractionnable sur une année. Sa prise en charge sera assurée par la sécurité sociale sur la base d'une indemnité journalière et complétée par l'employeur, pour garantir au salarié le maintien de son niveau de revenu. Les travailleurs indépendants bénéficieront d'un congé de quinze jours qui donnera droit à une indemnité journalière de la sécurité sociale. Quant à elle, la commission des lois du Sénat est à l'initiative d'un amendement, adopté en commission, visant à rétablir une équité de traitement entre les agents du secteur public et les salariés du secteur privé. En effet, la fonction publique d'État ne prévoit qu'un congé de trois jours pour les parents confrontés au deuil d'un enfant. Aussi, la commission propose un niveau de protection équivalent entre les secteurs public et privé. Pour reprendre les mots très justes de Philippe Bas, président de notre commission des lois, ces dispositions n'effaceront pas la douleur des parents, mais expriment la solidarité de la Nation face à ces épreuves. Le Gouvernement a également proposé un amendement ayant pour objet de prolonger, pour une durée de trois mois, le versement des prestations familiales aux familles confrontées à la perte d'un enfant. Enfin, notre collègue Catherine Deroche propose le versement d'une allocation forfaitaire de 2 000 euros afin de faciliter la prise en charge des frais d'obsèques. Financée par les caisses d'allocations familiales, cette allocation sera versée à toutes les familles concernées, sans conditions de ressources, mais elle sera modulable selon les revenus du foyer. Au nom du groupe Les Indépendants, je suis favorable à l'ensemble de ces dispositions adoptées en commission. Elles sont à la fois suffisamment protectrices pour aider au mieux chaque famille à traverser la terrible épreuve qu'est la perte d'un enfant et assez souples pour s'adapter aux situations personnelles de chacun.

pour examiner un important texte d'accompagnement de familles touchées par ce que chacun d'entre nous redoute : la perte d'un enfant. Je remercie Mmes les rapporteurs pour leur travail. Je remercie particulièrement Élisabeth Doineau d'avoir bien voulu intégrer, dès le début de la réflexion, la proposition de loi

Notre proposition de loi faisait suite à un travail mené depuis plusieurs années avec une association de notre département, l'Association Audrey, devenue Méningites France, engagée dans le soutien aux familles et dans la prévention des méningites, mais aussi des autres infections bactériennes ou virales. Je salue M. et Mme Voisine, qui sont présents dans la tribune, pour leur engagement sans faille depuis le décès de leur fille Audrey.

L'article 3 permet de considérer l'enfant à charge et de maintenir ainsi les prestations d'entretien pendant trois mois après le décès. L'article 4 crée une prestation forfaitaire pour faire face au décès d'un enfant mineur, notamment aux frais d'obsèques. Cette prestation sera versée sans conditions de ressources, mais avec un plafond fixé par décret et une modulation en fonction des ressources du foyer.

nous examinons, la période d'absence supplémentaire de huit jours peut être prise dans les douze mois suivant le décès. J'approuve cette souplesse apportée. En revanche, et nous allons en débattre, le terme de « répit » ne me satisfait pas pleinement. J'avais proposé deux autres dispositions : la première, à savoir la transmission automatique des actes d'état civil aux caisses d'allocations familiales est désormais satisfaite

Si la patience dont il est question est une sagesse, alors je veux croire que le Sénat, dans ce bicamérisme français, en fait notamment preuve lorsqu'il faut faire aboutir une proposition de loi. Mais surtout, s'il est des personnes dont le temps est compté- un temps devenu si précieux -, ce sont bien ces parents dont l'enfant est parti trop tôt, beaucoup trop tôt C'est tout le sens du message qu'a souhaité porter notre collègue député du groupe UDI, Agir et Indépendants, Guy Bricout, par son initiative. En effet, il faut du temps pour faire face à un tel drame, pour assumer les démarches administratives, pour préparer les obsèques et régler les formalités. Oui, il en faut pour accomplir, avec déchirement, les derniers devoirs de parents, ce qui, en cinq jours seulement, n'est pas toujours possible. Sans parler du temps de la douleur.

au nom même de cet élément temporel que je viens d'évoquer et pour affirmer, collectivement, un message de soutien rapide à ces parents. On nous dira que le texte initial n'était pas parfait, qu'il n'optait pas pour le bon financement ou qu'il devait peut-être s'inscrire dans une approche plus globale.

Un grand hebdomadaire indiquait qu'une députée de la majorité n'y avait pas pensé. Apparemment, elle ne devait pas être la seule, car, lors de la réunion interministérielle du 17 janvier dernier, le Gouvernement non plus n'a pas eu cette idée. Permettre à des parents frappés par le malheur, désorientés par le choc, parfois laissés dans le désarroi le plus profond, de bénéficier d'un peu plus de temps, voilà un sujet qui ne méritait pas la moindre polémique. Au lieu de cela, la majorité est revenue, en première lecture, sur la mesure phare de cette proposition de loi, en modifiant en commission la rédaction de l'unique article. C'est regrettable pour l'image que cela renvoie du débat parlementaire, pour l'incompréhension que cela a suscité chez les Français, pour des raisons de justice sociale, dans laquelle la République puise ses fondements. Devant vous, mes chers collègues, je l'affirme : la République, ce n'est pas un slogan ; c'est avant tout une force de conviction ! L'émotion a été grande dans tout le pays. Cette situation a beaucoup choqué. Nous pouvons d'ailleurs saluer le soutien public du Medef. Car, oui, les entreprises ne sont pas étrangères à la douleur de leurs salariés. Ainsi fallait-il attendre un tweet pour que, enfin, le texte suscite une attention nouvelle. Aussi, la proposition de loi arrivée au Sénat était totalement modifiée et comportait deux articles, bien en deçà des ambitions exprimées initialement.

Je tiens à saluer ma collègue Élisabeth Doineau, rapporteure, pour sa détermination qui a permis de compléter ce texte et de lui donner une envergure tout autre, ainsi que notre collègue Catherine Di Folco, rapporteure pour avis. Désormais, l'article 1 porte à sept jours ouvrés, à la charge de l'employeur, la durée du congé pour événement familial, en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Il crée également un congé de deuil d'une durée maximale de huit jours, pendant lesquels le salarié bénéficierait d'une indemnité journalière de la sécurité sociale. Ces huit jours d'absence seraient fractionnables et pourraient être pris dans l'année suivant le décès de l'enfant. Cette entraide privé-public est fondamentale, car la solidarité nationale a également un rôle à jouer. surtout, les fonctionnaires- sur ce point, mais aussi sur celui de l'autorisation spéciale d'absence-, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles sont pris en compte. Je ne reviendrai pas sur les détails techniques de ces dispositions ou de celles qui tendent à tenir systématiquement compte de l'enfant décédé dans le calcul du RSA. RSA. Il s'agit de points majeurs qui permettent à ce texte d'être le plus complet possible. En outre, une question a été soulevée par notre collègue Catherine Deroche, qui a d'ailleurs été à l'initiative d'une belle proposition de loi portant diverses mesures d'accompagnement des parents en cas de décès d'un enfant mineur, mineur, sur le maintien des prestations familiales durant les trois mois suivant le décès de l'enfant. Cette proposition de loi consacre désormais ce droit pour les prestations générales d'entretien de l'enfant- seraient ainsi concernées, par exemple, les allocations familiales et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. handicapé. L'enfant décédé sera donc considéré, pendant cette période, à la charge effective et permanente de la famille pour apprécier les conditions d'attribution de l'ensemble des prestations servies au foyer, au titre d'un autre enfant- comme l'allocation de rentrée scolaire versée à un autre enfant. Le enfant. Le choix a été fait d'apporter une mesure de protection contre le licenciement, durant un délai de treize semaines. Si elle peut permettre de favoriser une protection optimale du salarié, alors nous la soutenons. concerne la question du don de RTT, l'article 2 a été réécrit substantiellement. Je salue le fait que ce dispositif de solidarité soit étendu aux agents publics. plus, afin de soutenir le revenu des familles endeuillées pendant une période d'exceptionnelle fragilité, la commission a décidé de supprimer le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant dans un délai de treize semaines à compter du décès de l'enfant. Cette mesure, applicable également aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants, s'inscrit dans le bon sens. Nous le savons, les frais d'obsèques sont très onéreux. Permettre aux parents d'acquitter les frais d'obsèques grâce à une nouvelle allocation forfaitaire, modulée selon les conditions de ressources, c'est le témoignage de la Nation tout entière à ses enfants. Surtout, c'est un point auquel j'accorde une très grande importance, il est vital que cette solidarité puisse s'exprimer au travers d'un accompagnement psychologique des parents et des frères et soeurs. Je salue la mise en place de cette expérimentation. Le choc émotionnel ne saurait être exprimé par mes simples mots, tant la situation peut être bouleversante pour une famille entière. Mes chers collègues, madame la ministre, la démocratie sort grandie de faire progresser les droits sociaux pour une République qui rassemble, pour une République plus juste, pour une République fidèle à ses valeurs. Pour toutes ces raisons, et saluant de nouveau ce travail de collaboration entre le Sénat et le Gouvernement, le groupe Union Centriste votera favorablement ce texte. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la perte d'un enfant est la plus douloureuse épreuve que peut rencontrer un parent dans la vie, parce que c'est un deuil contre nature. Pour y faire face, les salariés disposent actuellement d'un congé de cinq jours, pris en charge par leur employeur. Cette durée est nettement insuffisante pour couvrir les nombreuses démarches nécessaires aux obsèques de l'enfant et permettre aux parents de se relever. Les salariés concernés n'ont alors pas d'autre solution que de prendre des congés décomptés sur leurs vacances ou de demander un arrêt maladie. dernier cas, les trois jours de carence s'appliquent, avec les conséquences financières induises. Au final, les parents qui font face à la perte d'un enfant restent peu soutenus par les pouvoirs publics. La proposition de loi de notre collègue député, M. Bricout, vise à remédier à cette situation en étendant la durée du congé à douze jours ouvrables en cas de décès d'un enfant mineur, ou à charge, au sens du droit de la sécurité sociale. En effet, les parents endeuillés ne sont généralement pas en mesure de reprendre leur travail à l'issue des cinq jours prévus dans le code du travail. Face au deuil d'un enfant, les parents prennent en moyenne trente-cinq jours d'arrêt maladie. La durée de cinq jours actuellement en vigueur est bien inférieure à celle qui est appliquée au Royaume-Uni, où, depuis l'adoption du, certains salariés peuvent bénéficier de deux semaines de congé de deuil pendant lesquelles ils sont rémunérés. L'employeur a l'obligation de verser à son employé sa rémunération habituelle. Ces jours peuvent être pris de manière discontinue. En Suède, la loi autorise un congé parental de dix jours pendant lequel la sécurité sociale prend en charge la rémunération du salarié. le décès d'un enfant a fait l'objet de débats houleux à l'Assemblée nationale. Les députés du groupe La République En Marche ont vidé le texte de sa substance. Je tiens à vous faire part de mon indignation en tant qu'élue, en tant que médecin et en tant que mère. Évidemment qu'on ne peut pas déterminer le deuil d'un enfant en nombre de jours ! Mais cette proposition de loi est une façon de reconnaître les souffrances de ces parents et de ces familles ; au-delà des parents endeuillés, il y a parfois des frères et des soeurs qui ont aussi besoin que leurs parents s'occupent d'eux. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, à condition qu'un accord collectif l'autorise, que le salarié pourra prendre tout ou partie des jours de congés annuels ou de RTT dont il dispose au moment de la perte d'un enfant. Mais les congés payés ne sont pas faits pour permettre aux salariés de se remettre du décès d'un enfant. Cette position est incompréhensible. La seule évolution, mesquinement consentie par les députés En Marche, est l'impossibilité pour l'impossibilité pour l'employeur de s'opposer, dans le meilleur des cas, à ce que le salarié prenne ses congés annuels à la suite de son congé de deuil. C'est donc à la Haute Assemblée qu'il revient d'humaniser ce texte, avec le soutien du Gouvernement qui consent désormais à reconnaître le manque d'humanité de la version votée par les députés de la majorité. La commission des affaires sociales a su faire preuve de compassion. Elle a augmenté la durée du congé pour événement familial, rémunéré par l'employeur, à sept jours ouvrés en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Une période d'absence supplémentaire de huit jours en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans a été créée, portant ainsi le total des droits d'absence des salariés concernés à quinze jours. Cette autorisation d'absence, appelée pour l'instant « congé de répit », pourra être prise séparément du congé pour événement familial dans le délai de douze mois suivant le décès. À la différence du congé pour événement familial, la rémunération de ces huit jours d'absence pourra être partiellement prise en charge par la solidarité nationale. En pratique, le salaire sera maintenu par l'employeur et fera l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale sous la forme d'indemnités journalières. En commission des affaires sociales, nous avons étendu ce congé aux travailleurs indépendants et aux agents publics. Le texte prévoit également le maintien des droits aux prestations familiales pendant un délai déterminé après le décès d'un enfant, ainsi que le maintien de la prise en compte de l'enfant au titre des droits au RSA. Enfin, à la suite de l'adoption d'un amendement de ma collègue Catherine Deroche, ce texte crée une allocation forfaitaire versée automatiquement aux familles en cas de décès d'un enfant à charge. Je tiens à saluer le travail remarquable des rapporteurs Élisabeth Doineau et Catherine Di Folco, ainsi que celui des associations qui soutiennent les familles endeuillées. Le Sénat s'honore d'avoir fait preuve d'humanité et de fraternité.

le congé de deuil pour les parents confrontés à la mort de leur enfant, la majorité a démontré, s'il en était encore besoin, son entêtement et une absence totale de sens politique face à un texte qui aurait dû emporter l'adhésion de tous. Plus grave encore, le compte rendu des débats révèle aussi le degré de dysfonctionnement et d'amateurisme du Gouvernement, qui aurait pu, en déposant un amendement, transférer la charge financière des entreprises à la solidarité nationale. La polémique aurait ainsi été largement évitée. De même, le texte adopté était complètement inadapté à la situation des petites entreprises, des artisans et indépendants, ou à la fonction publique.

La polémique a ensuite donné lieu à une véritable surenchère, à la fois dans les déclarations du Président de la République, qui demandait de faire preuve d'humanité, et de la majorité. Le Gouvernement a ensuite souhaité apparaître comme le plus donnant, en proposant notamment un plan global d'accompagnement des familles endeuillées. Alors, après avoir refusé les douze jours, on passait à quinze ... Et pourquoi pas davantage ? Quel que soit le nombre de jours donnés, il est bien évident que la douleur des familles ne s'éteindra jamais. Attention donc à ne pas tomber dans une sorte de contagion des émotions. En commission des affaires sociales, nous avons examiné plusieurs amendements du Gouvernement reprenant, pour une large part, les dispositions contenues dans une proposition de loi déposée en juillet 2019 par notre collègue Catherine Deroche et collant, là aussi, aux propositions de notre rapporteure Élisabeth Doineau- preuve, s'il en était besoin, que le Sénat n'est pas déconnecté des préoccupations et des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens. Les dispositions votées en commission me semblent en effet répondre à une réelle demande des parents endeuillés, notamment l'allongement à sept jours du congé actuellement prévu par le code du travail et pris en charge par l'employeur et la création d'un congé de deuil supplémentaire de huit jours pris en charge, pour partie, par la sécurité sociale. Mais cessons de parler de « congé de répit ». De répit, il n'y en aura plus jamais pour ces parents. Il s'agit d'un congé de deuil, et rien d'autre. Permettez-moi, cependant, d'émettre quelques réserves sur le fait que ce congé soit fractionnable et qu'il puisse être pris plus tard dans l'année suivant le décès de l'enfant.

Enfin, et surtout, il me paraissait très important d'étendre à l'ensemble des actifs, salariés du secteur privé, mais aussi travailleurs indépendants et agents publics, le nouveau dispositif.

Darcos, sur l'article. Permettez-moi de saluer ici le travail remarquable d'humanité accompli par la commission des affaires sociales, lequel contraste singulièrement avec la première approche de l'Assemblée nationale. La disparition d'un enfant est une tragédie. Parce qu'elle n'est pas dans l'ordre des choses. Parce que la logique voudrait que l'adulte s'en aille avant l'enfant, qui a tout l'avenir devant lui. Quelle qu'en soit la cause, accidentelle ou conséquence d'une maladie, elle laisse les familles dévastées. À cet instant, je ne peux m'empêcher d'évoquer l'écrivain Philippe Forest : dans une tribune publiée récemment dans le journal, il relate avec une pudeur mêlée d'une douleur incommensurable la perte de sa petite Pauline, décédée d'un cancer à l'âge de 5 ans. L'écrivain considère que, si le « deuil d'un enfant est et restera toujours intolérable », le débat sur le nombre de jours de congé qu'il convient d'accorder aux parents en deuil, certes dérisoire, n'en est pas moins nécessaire. C'est pour lui un « signe salutaire » que la Nation adresse à celui qui est privé d'enfant et « par lequel elle prend acte, autant qu'elle le peut et sans être en mesure de la soulager pourtant, de l'épreuve qu'il traverse Dans ce contexte, l'allongement du congé pour événement familial de cinq à sept jours et la création d'un congé de répit d'une durée maximale de huit jours sont de nature à répondre, en partie, à la situation des familles endeuillées. Ces dernières ont besoin de temps pour s'organiser matériellement et pour essayer de se résoudre à l'absence de l'être cher, si tant est que l'on puisse un jour s'y habituer. Si je souhaite prendre la parole sur cet article, c'est également pour évoquer un drame que cette proposition de loi ne prend pas en compte, celui de la mort intra-utérine d'un enfant. Tout aussi violente, tout aussi douloureuse que celle d'un enfant né vivant. Pour la femme qui a porté l'enfant, pour le couple qui préparait sa venue, le drame est immense et le deuil, le temps du deuil, n'en est pas moins nécessaire. Pourquoi ne pas étendre ces droits à congé et au répit aux parents concernés ? Je regrette sincèrement de ne pas en avoir parlé plus tôt avec mes collègues de la commission des affaires sociales. De même serait-il judicieux, de mon point de vue, d'élargir ultérieurement aux parents, frères et soeurs d'un enfant mort-né le droit à une prise en charge psychologique des familles endeuillées, tel que le prévoit l'article 6 de la proposition de loi, du moins à titre expérimental dans un premier temps. Je souhaite que le Gouvernement ouvre une réflexion sur le sujet. Dans cette attente, je demande à l'assurance maladie un peu plus de compassion quand elle informe les parents d'enfants décédés avant la naissance qu'ils ne peuvent bénéficier du droit à l'indemnisation de leur congé maternité. La

Cet article, qui corrige l'erreur initiale, est plus conforme à l'esprit de solidarité et d'accompagnement des parents en deuil en améliorant les droits d'absence des salariés à la suite du décès d'un enfant. Ces modifications sont bienvenues. Qu'elles soient le fruit d'une négociation avec le Gouvernement était nécessaire pour sortir par le haut de l'erreur d'appréciation dans laquelle s'était fourvoyée l'Assemblée nationale, obstinée et s'enfermant dans une argumentation technique. Pour autant, il n'y a pas lieu de faire un concours de pathos et de surenchérir dans l'ostentation d'humanité. Si je me réjouis de ce changement d'attitude et du fait que le Gouvernement se soit racheté en réparant son erreur initiale, je retiendrai deux choses de cet épisode malheureux que nous réparons aujourd'hui. D'abord, en dépit de ce changement de pied du Gouvernement et des dispositions plus favorables pour mieux accompagner les familles qui ont perdu un enfant, la mort d'un enfant reste la mort d'un enfant, c'est-à-dire une expérience incommensurable et, dans une large mesure, indicible. Aucune disposition législative ne saurait véritablement soulager la douleur de la perte d'un enfant et il appartiendra à chacune des familles de décider si elle souhaite bénéficier ou non de ce congé supplémentaire. Le second enseignement est d'un niveau bien différent et porte sur la conception un peu trop exclusive que se fait le Gouvernement du travail législatif. Il ferait mieux, je pense, de s'interroger sur les conditions d'élaboration de la loi et de reconsidérer sa propension un peu trop naturelle à légiférer de manière unilatérale et exclusive.

Lors des débats en commission, la question s'est posée des personnes- salariés, travailleurs indépendants, demandeurs d'emploi ou fonctionnaires -confrontées au deuil d'un enfant ou d'un jeune de moins de 25 ans, ne disposant pas d'un lien de filiation directe avec l'enfant décédé, mais en assumant la charge effective. s'agit d'une question importante qui a fait l'objet de plusieurs amendements, notamment de la part de Mme Di Folco. Toutefois, certains de ces amendements n'étaient pas recevables au titre de l'article 40 nous partageons totalement l'idée que ce congé, comme l'ensemble des droits nouveaux créés par cette proposition de loi, doit être ouvert aux personnes qui assument la charge effective de jeunes de moins de 25 qui

également d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Cette disposition permet ainsi de tenir compte de différentes situations, par exemple dans le cas des familles recomposées, et d'inclure les enfants qui, sans avoir de filiation directe, étaient à la charge du salarié.

: La parole est à Mme Catherine Di Folco. Les mots ont un sens. Il me paraît fondamental de les utiliser à bon escient. Quelle est la définition du mot « répit » ? C'est la suspension de quelque chose de pénible, d'une souffrance. Quelle est la définition du mot « deuil » ? C'est la perte, le décès d'un parent. C'est une douleur, une affliction éprouvée à la suite du décès de quelqu'un. Les synonymes de deuil sont affliction, chagrin, déchirement, malheur, épreuve Pour affronter une épreuve, il faut la regarder en face et, pour cela, la nommer justement. Le deuil n'est pas un état de fatigue ou quelque chose de pénible que l'on peut suspendre. C'est un déchirement, une blessure qui ne peut cicatriser et avec laquelle il faut réapprendre à vivre.

J'avais 14 ans ; mon petit frère 11 ans ; ma petite soeur 7 ans. Nous avons largement apprécié la présence de notre grand-mère pour soutenir notre père.

les familles endeuillées. Cet amendement revient à l'esprit initial de la proposition de loi, en étendant ce dispositif au décès d'un enfant à charge. Cette notion permet d'inclure les enfants qui, sans avoir de filiation directe avec les agents publics, sont à leur charge. Elle est particulièrement importante pour les familles recomposées, car elle ouvre ce droit aux enfants du conjoint, partenaire de PACS ou

Di Folco. Cet amendement encourage le don de jours de repos dans la fonction publique en simplifiant les procédures. Ce don est strictement encadré, dans l'objectif de préserver la santé des agents. À titre d'exemple, leurs jours de récupération et leurs vingt premiers jours de congés payés ne peuvent pas être « transférés » à un collègue. Les agents « donateurs » doivent également obtenir l'accord de leur chef de service. Cette règle paraît superfétatoire : sans remettre en cause le bon fonctionnement du service, il est proposé de la remplacer par une simple obligation d'information.

Mme Catherine Di Folco. De manière opportune, l'article 7 prévoit que le contrat de travail d'un salarié ne peut pas être rompu pendant les treize semaines suivant le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d'étendre cette règle aux agents contractuels de droit public. Revenant à l'esprit initial de la proposition de loi, cet amendement permet d'inclure au dispositif les enfants qui, sans avoir de filiation directe avec les personnes concernées, sont à leur charge. Il vise en particulier, comme précédemment, les enfants du conjoint, partenaire de PACS ou concubin dans les familles recomposées. Comme c'est la dernière fois que je prends la parole sur ce texte,

qui correspond, en réalité, au niveau maximal pouvant être attribué par les caisses d'allocations familiales sur le territoire. En effet, au travers du droit

nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP). Ce texte, que je vous présente cet après-midi avec Agnès Pannier-Runacher, vient marquer une nouvelle étape dans la transformation de l'action publique. l'initiative du Président de la République, le Gouvernement a engagé l'année dernière un grand débat national permettant à toutes et à tous de débattre des questions essentielles pour les Français. Les contributions ont fait émerger une demande forte de transparence, de proximité et de simplification dans les relations entre les citoyens et l'administration.

Afin de répondre aux attentes fortes de nos concitoyens, le Gouvernement entend accélérer la dynamique en matière de simplification et d'efficacité administratives, à travers plusieurs mesures très concrètes. L'objet des seize premiers articles du titre I de ce texte est ainsi de simplifier le paysage administratif,

remise dès 2007 d'un rapport d'information sur la suppression des commissions et instances consultatives placées auprès du Premier ministre ou par la création en 2018 d'un « bureau d'abrogation des lois anciennes inutiles », le Sénat a toujours fait preuve d'une rigueur en la matière. Dans ce même esprit de rationalisation, le Gouvernement souhaite aujourd'hui la suppression ou le regroupement thématique de certaines commissions, afin de faire disparaître des consultations à la portée limitée, de fluidifier la décision publique et de mobiliser des agents sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour les Français.

la commission spéciale a apporté des modifications substantielles au texte, en refusant notamment la disparition ou le regroupement de certaines commissions, comme l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement ou le Conseil supérieur de la mutualité.

Cela me donnera aussi l'occasion de vous apporter plus d'explications concernant l'objectif du Gouvernement sur ces différentes thématiques et les raisons qui nous avaient conduits à proposer la suppression de tel ou tel organisme. Le nombre important de ces structures à la configuration et au statut juridique variés nuit à la lisibilité de l'administration pour les usagers

le Gouvernement a été particulièrement sensible aux arguments avancés par les sénateurs en commission spéciale et a décidé de suivre votre avis. Par conséquent, nous ne proposerons pas le rétablissement de cet article. De plus, un amendement gouvernemental De plus, un amendement gouvernemental visera à intégrer dans le corps législatif la nouvelle politique d'indemnisation mise en oeuvre par le Comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires (Civen). Palliant l'absence de dispositions transitoires, cette politique de reconnaissance augmentera le nombre des bénéficiaires d'une indemnisation et améliorera ainsi le système de prise en charge des victimes.

à insérer un article additionnel tendant à réviser la périodicité du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, pour la porter de trois à cinq ans. La dimension stratégique de ce plan sera renforcée par la mise en cohérence avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui intervient elle aussi tous les cinq ans. Si cet amendement

Nous nous sommes fixé l'objectif de rapprocher 99 % des décisions individuelles des acteurs concernés afin de répondre à la double attente de proximité et de rééquilibrage des institutions et des structures économiques sur l'ensemble du territoire. Ainsi, le titre II du projet de loi a pour objet de déconcentrer les décisions administratives individuelles. Cette prise de décision au niveau le plus adapté permettra de renforcer le lien entre les administrations et les usagers des services publics. réjouis, là encore, qu'une grande partie de ces mesures de déconcentration aient reçu un accueil favorable de la part de la commission spéciale. Eu égard aux contraintes opérationnelles du terrain, plusieurs types de décisions seront ainsi déconcentrés. À titre d'exemples, le transfert au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) des décisions d'interdiction de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention

la délivrance des certificats de conformité aux bonnes pratiques des laboratoires par une seule et même autorité, le Comité français d'accréditation. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi témoigne de l'ambition du Gouvernement de renforcer les liens entre l'administration et les usagers,

tout d'abord simplifier la délivrance de divers documents, comme les papiers d'identité, le permis de conduire ou le titre de séjour, grâce à un dispositif dispensant, sous certaines conditions, de présenter un justificatif de domicile. Ensuite, nous voulons simplifier les démarches qui concernent nos jeunes concitoyens. Par exemple, l'inscription à l'examen du permis de conduire sera facilitée par la mise en oeuvre d'une plateforme en ligne où les places seront attribuées sans quotas ni classement selon l'ordre d'inscription.

plus proche de celle du texte initial. D'autre part, le projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises. Le Gouvernement souhaite rendre les procédures administratives plus efficaces et plus rapides, tout en maintenant nos exigences en matière d'urbanisme, d'archéologie ou d'environnement. Ces articles s'appuient sur la mission du député Guillaume Kasbarian, qui a analysé des cas réels de projets dont les promoteurs ont rencontré des difficultés pour s'implanter en France

Nous proposons de renforcer la sécurisation des porteurs de projet face aux changements réglementaires en cours de procédure. Les projets en cours d'instruction seront considérés comme des sites industriels existants, existants, soumis à toute nouvelle réglementation dans les mêmes conditions et délais d'entrée en vigueur. En revanche, il ne sera plus nécessaire de reprendre de zéro l'instruction d'un dossier. Nous souhaitons également faciliter l'instruction des dossiers en permettant aux préfets d'adapter les procédures aux situations particulières des territoires et des projets. Plusieurs autres mesures des titres IV et V visent également à simplifier la vie des entreprises. Je n'en citerai que certaines. En réponse En réponse aux demandes des organisations professionnelles et en accord avec les organisations syndicales, nous proposons de simplifier l'adoption d'accords d'intéressement une décision unilatérale de l'employeur dans les TPE, et partant de revenir à la rédaction initiale en concertation avec les pharmaciens, simplifier les formalités de vente en ligne de médicaments, en passant d'un régime d'autorisation à un régime déclaratif et en revoyant les règles qui régissent le nombre de pharmaciens devant être employés dans une officine en fonction de l'activité de cette dernière et non pas du chiffre d'affaires,

Le texte permet aussi certaines surtranspositions que vous connaissez bien pour les avoir votées en décembre 2018. Enfin, certains dispositifs touchent directement au quotidien de nos concitoyens, même s'il agit de questions apparemment techniques.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi est une réponse aux attentes nombreuses et diverses des Français quant à la nécessaire transformation de l'action administrative : il s'agit de décider plus vite, plus simplement, plus clairement, au plus près de nos concitoyens. Ces mesures doivent permettre un service public plus proche,

Monsieur le président, madame, monsieur les secrétaires d'État, mes chers collègues, le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique dont nous entamons la discussion s'inscrit dans une longue série de textes ayant pour objet la modernisation de l'administration et l'amélioration de son efficacité. Plus précisément, il répond à trois engagements pris par le Gouvernement l'administration plus simple, d'où la proposition de supprimer des commissions consultatives jugées inutiles, plus proche des Français, par la déconcentration des décisions, plus efficace et plus rapide, grâce à la modernisation et à la simplification des démarches courantes. Le Sénat s'est toujours exprimé positivement sur les dispositions des projets et des propositions de loi visant à améliorer l'efficacité de notre administration. Il en est de même de la commission spéciale : elle approuve toutes les mesures ayant pour objet de simplifier les normes et les procédures qui entravent inutilement les initiatives des particuliers ou des entreprises, et en conséquence le développement économique et l'emploi. Nous avons donc examiné avec bienveillance et sans négatif les propositions gouvernementales de suppression ou de fusion de commissions administratives consultatives, au nombre de quinze au total. Le Gouvernement justifie ces propositions par plusieurs motifs l'absence d'activité de ces commissions, leur caractère superfétatoire en raison de l'existence d'autres organismes similaires, enfin leur coût de fonctionnement et la perte de temps administratif au détriment d'actions à plus forte valeur ajoutée pour nos concitoyens. La commission spéciale a toutefois procédé à un examen approfondi de l'activité et des domaines de compétence de ces commissions. Elle a constaté que certaines avaient une activité soutenue, un rôle déterminant pour l'information des citoyens et la transparence de l'action publique ou assuraient une fonction de recours indispensable en cas de désaccord ou de contestation des niveaux de concertation inférieurs. inférieurs. En conséquence, elle a refusé la suppression de plusieurs de ces commissions ou adopté des dispositifs évitant leur disparition « sèche Pour ce qui concerne la déconcentration de certaines procédures et de la prise de décisions administratives individuelles dans les domaines de la culture, de la propriété intellectuelle et de la santé, qui vise à transférer à des organismes administratifs déconcentrés la prise de décision formellement assurée par les ministres concernés alors que les organismes en assuraient l'instruction, la commission spéciale a considéré qu'il s'agissait d'une mesure bienvenue d'allégement des procédures. elle a exclu de cette évolution la question très sensible des labels de la création artistique, compte tenu des enjeux en matière d'aménagement culturel du territoire et d'égalité territoriale dans l'accès à la culture. Elle a approuvé également les mesures de simplification administrative proposées concernant surtout des procédures obsolètes, les suites d'expérimentations abouties ou des dispositions d'ajustement des textes en vigueur.

entre exigence de défense de l'environnement et besoins de la vie économique. Elle n'y a apporté que des précisions rédactionnelles. Toutefois, le Gouvernement ne s'en est pas tenu à ces mesures qui justifiaient l'intitulé

un texte d'un genre que nous n'apprécions pas, ici au Sénat, car source de beaucoup de frustrations, aucun sujet ne pouvant être correctement traité dans son contexte et dans toutes ses implications.

l'irrecevabilité des cavaliers législatifs ou parce que la navette parlementaire a été abandonnée en raison de l'encombrement de l'ordre du jour du Parlement. La commission spéciale n'est bien sûr pas opposée à ces mesures ; elle a même profité de l'occasion pour réintroduire dans le processus législatif de navette avec l'Assemblée nationale des avancées votées par la Haute Assemblée et favorables aux droits des citoyens consommateurs et à l'information des élus locaux ou destinées à améliorer les processus administratifs. Je pense par exemple à la simplification de l'approvisionnement en médicaments des officines ou à la clarification des modalités d'application du droit de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur. ne sont pas mauvaises sur le fond, mais elles illustrent les difficultés que nous rencontrons pour débattre sereinement dans de bonnes conditions, puisque nous sommes contraints à des repentirs et à des ajustements très rapides après le vote d'une loi. loi. Surtout, ce projet de loi contient des mesures qui n'ont qu'un lointain rapport avec la simplification de l'action publique et dont certaines sont très contestées par les acteurs des secteurs d'activité concernés- je pense évidemment aux avocats et aux pharmaciens. Ces articles nous ont donné le sentiment d'avoir été raccrochés au texte sans préparation suffisante, surtout parce que celui-ci constituait un véhicule législatif commode dans un agenda législatif surchargé. Ces dispositions très contestables, dont certaines ont un caractère quasiment provocateur, concernent des thèmes variés. Le service national universel, par exemple, qui n'a jamais été débattu au Parlement, est abordé sous l'angle bien étroit d'une habilitation à légiférer par ordonnance sur le recrutement des encadrants. Elles concernent aussi les seuils de revente à perte et les promotions pour les denrées et certains produits alimentaires ou les règles applicables aux personnels de l'Office national des forêts et à son conseil d'administration, deux questions sur lesquelles le Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance, sans manifestement avoir tenu compte des travaux parlementaires. Sur tous ces sujets, la commission spéciale estime qu'un vrai débat doit avoir lieu et elle ne souhaite pas donner carte blanche au Gouvernement. Enfin, au nom de la commission spéciale, je regrette que l'examen du projet de loi se déroule dans des conditions assez acrobatiques. Absolument ! D'abord, les délais sont particulièrement brefs, ce qui m'a contrainte à limiter le nombre et la durée des auditions.

est sans doute un voeu pieux, puisque la nature des amendements déposés en dernière minute par le Gouvernement, que nous avons écartés au titre de l'irrecevabilité des cavaliers législatifs

à la fin du titre II et avant le titre III, soit entre les articles 20 et 21. du Gouvernement pour que l'article 33, ainsi que les amendements portant articles additionnels après l'article 33, soient examinés en priorité à la fin du titre II. Quel est l'avis de la commission spéciale sur cette demande de priorité formulée

Néanmoins, nous ne pouvons que critiquer la méthode choisie pour l'examen de ce texte. Un mois à peine s'est écoulé entre sa présentation en conseil des ministres et son examen en séance : c'est fort peu pour mesurer toutes les implications et les incidences d'un texte qui compte près de cinquante articles touchant aux sujets les plus divers, les plus complexes et les plus techniques. Finalement, l'acronyme par lequel on « simplifie » son titre présente le mérite de la clarté quant à l'objectif du Gouvernement

Je tiens donc à saluer les travaux de la commission spéciale chargée d'examiner ce projet de loi et particulièrement de sa rapporteure, Patricia Morhet-Richaud, qui a rempli sa mission en un temps record et a permis de faire évoluer le texte en partie dans le bon sens. Les sénateurs socialistes y ont pris toute leur part. Dans un esprit constructif, et parce que des dispositions allaient dans le sens d'une réelle simplification, nous avons, en accord avec la commission spéciale, approuvé ou simplement précisé près de la moitié des articles de ce texte. Mais d'autres mesures ne sont pas du tout anodines et n'ont que peu de rapport avec la simplification de l'action publique. La commission spéciale les a modifiées ou supprimées. Ainsi, je me félicite du maintien de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires. Monsieur le secrétaire d'État, vous l'avez reconnu vous-même : comment pouvait-on envisager la suppression de cette commission, alors que votre objectif est le démantèlement de quatorze réacteurs d'ici à Je me félicite également du remplacement de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur l'expérimentation de l'encadrement des promotions et du relèvement des seuils de revente pour les denrées et certains produits alimentaires par une prorogation sous conditions. La commission aménage ainsi certains dispositifs problématiques de la loi Égalim et de cette ordonnance, que nous avions fortement mis en exergue dans le cadre d'une mission d'information De même, nous avons demandé et approuvé la modification des dispositions concernant les avocats et les pharmaciens. En effet, en supprimant la possibilité de vente de médicaments par des plateformes en ligne et celle d'exercer cette activité en stockant dans des locaux distincts des officines, nous avons évité une certaine forme d'« ubérisation » de la santé. Enfin, l'autorisation, pour l'assureur de protection juridique, d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et son avocat était préjudiciable à cette profession et à ses clients ; nous l'avons donc supprimée.

la mise en place, sur proposition de notre groupe, d'antennes de pharmacie pour préserver l'accès à une offre pharmaceutique dans les communes isolées, à des mesures de simplification en matière de résiliation d'un contrat assurance emprunteur, qui reprennent la proposition de loi socialiste de Martial Bourquin adoptée à l'unanimité au Sénat en novembre dernier. Cependant, ces modifications auraient pu aller encore plus loin, s'agissant particulièrement des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que du maintien de la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'État outre-mer- je suis certaine que nos collègues ultramarins y reviendront -et de la suppression du recours à la simple consultation du public pour certains projets soumis

Un sujet de cette importance ne saurait être traité de cette façon. La gestion de notre forêt et l'avenir de l'ONF doivent faire l'objet d'un débat et d'une réforme à part entière. Je suis au regret de devoir vous dire que, selon nous, votre réponse au grand débat national ne répond pas aux préoccupations des Français. Bien au contraire, certaines de vos « simplifications » leur envoient un très mauvais signal. Ils demandent des services publics plus lisibles, plus proches et plus accessibles dans tous les territoires, sans exception. Or suppression n'a pas valeur de simplification : c'est l'aveu d'un manque de réflexion et de l'absence totale d'un véritable projet politique que de le croire. Les avancées obtenues en commission sont heureuses, mais encore insuffisantes, et je souhaite que nos débats en séance publique puissent nous permettre d'obtenir de nouvelles garanties sur tous les sujets que j'ai évoqués et qui restent en suspens. La parole

simplifier, déconcentrer et supprimer : tels sont les trois maîtres mots du projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui. L'objet est louable, dans une période où nos concitoyens aspirent à davantage de fluidité et de rapidité dans leurs rapports avec l'administration,

qui a su revenir sur certaines dispositions pouvant paraître inopportunes, relatives notamment, au titre I, à la suppression de certaines commissions administratives. J'entends qu'il qu'il faille supprimer bon nombre de commissions dont l'utilité n'a pas été prouvée, mais, comme pour tout, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, au risque de s'égarer en chemin.

Pour en revenir au présent texte, j'approuve les modifications introduites à l'article 8 par la commission spéciale. Elles permettent de maintenir la participation des élus locaux et des associations oeuvrant dans les domaines du logement et de l'insertion aux débats du futur haut comité pour le logement des personnes défavorisées et pour le suivi du droit au logement opposable.

concerne les mesures de déconcentration de la prise des décisions administratives dans les domaines de la culture et de la santé, je retiens le transfert au directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament de la liste des médicaments pouvant être rétrocédés.

Le risque, à moyen et long termes, aurait été de fragiliser l'activité des officines de petite taille et de mettre à mal des commerces de proximité qui n'ont pas besoin de cela. de cela. Enfin, je relève l'assouplissement des conditions de recrutement des pharmaciens adjoints. Sera prise en compte la marge réalisée par les pharmaciens, et non plus uniquement leur chiffre d'affaires.

L'équilibre entre nécessité d'accélération des procédures, protection de l'environnement et information des parties concernées est plutôt respecté. Je pense à l'article Je pense à l'article 25, qui introduit un droit d'information du maire sur les projets d'installation d'éoliennes avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale ou aux mesures assimilant les dossiers en cours d'instruction à des ICPE existantes.

il serait nécessaire de simplifier les démarches pour l'accès aux différentes prestations sociales. Quand on sait que, pour certaines aides, le taux de non-recours atteint 40 %, il y a de quoi s'interroger.

La loi Essoc « pour un État au service d'une société de confiance » a marqué une première étape, avec le principe du « dites-le-nous une fois », la création d'un droit à l'erreur, la dématérialisation de toutes les démarches avec l'administration, ou encore la fin des numéros surtaxés pour joindre les administrations et services de l'État.

La loi de transformation de la fonction publique a également apporté de nouveaux outils au service de la simplification de l'action administrative : les missions des commissions administratives paritaires sont recentrées sur le champ disciplinaire

Dans ce cadre de simplification de l'organisation administrative, le titre I du projet de loi prévoit la suppression d'un certain nombre de commissions consultatives. On compte encore 396 comités Théodule ; 86 d'entre eux seront supprimés. Il s'agit Il s'agit de réduire les doublons avec d'autres organes de consultation, de supprimer des commissions qui ne se réunissent plus, mais aussi de privilégier d'autres modes de consultation, moins administratifs et plus ouverts sur la société : l'essentiel, c'est ce qui est utile, ce que sentent, ce que veulent les Français.

Cela ne signifie pas- je le dis avec d'autant plus d'assurance que je soutiens, bien entendu, l'initiative du Gouvernement -que le Parlement ne doive pas être informé sans aucune ombre sur les conséquences de ces suppressions

troisième bloc de mesures que contient ce projet de loi a trait à la simplification des démarches pour les Français et pour les entreprises. Je l'ai dit en dressant un parallèle avec la loi Essoc

l'une des « mesures pour un permis pour tous, moins cher et plus rapide » présentées par le Premier ministre en mai 2019. Dans les territoires ruraux, nous savons les difficultés liées à l'obtention du permis de conduire. Combien de jeunes refusent un emploi parce que les transports en commun sont structurellement insuffisants ?

à mon tour : ce projet de loi compte un grand nombre de mesures, parfois très lourdes, sur des sujets appelant une évaluation des politiques actuelles et la construction d'une stratégie transparente. Compte tenu des délais resserrés pour l'examen du membres de notre groupe déplorent eux aussi, la navette parlementaire devra permettre de circonscrire ou d'enrichir le texte. La commission spéciale du Sénat y a toutefois déjà utilement contribué. Je pense

En Marche voteront ce texte. Nous saluons tant le travail du Gouvernement que celui de notre assemblée pour rendre la vie des Français, usagers des services publics ou entreprises, plus simple

Le triptyque accélération-simplification-modernisation devient une sorte de laissez-passer, de sésame justifiant le retrait de l'État et une perte de compétences de l'administration centrale, le recul de procédures protectrices, en particulier en droit de l'environnement, la disparition pure et simple de certaines commissions ayant le mérite d'apporter une analyse critique indépendante de certaines politiques publiques et d'informer nos concitoyens, nos concitoyens, la déconcentration de certaines décisions administratives individuelles sensibles, qui risque de placer les autorités déconcentrées en situation de conflit d'intérêts, ou encore- nous y reviendrons -la privatisation de l'ONF et la remise en cause de modes d'accueil de la petite enfance. Pis, ce sésame permet au Gouvernement

Enfin, comme le souligne justement Mme la rapporteure, « l'administration s'est trop souvent révélée incapable de fournir les informations demandées, notamment sur les dispositions des ordonnances pour lesquelles une habilitation est demandée par le Gouvernement

des plateformes de vente en ligne de médicaments, par la privatisation de l'ONF et du réseau des chambres d'agriculture, par la remise en cause du service universel du permis de conduire et du service national universel, par la privatisation rampante et la destruction des structures d'accueil de la petite enfance.

les restructurations des services administratifs s'intensifient avec la réduction des personnels, la mutualisation des fonctions et la privatisation de certains services. Ce sont autant de moyens directs ou indirects en moins pour accompagner les entreprises et les particuliers dans l'ensemble des territoires. C'est pourquoi nous pensons que l'étendard brandi de la simplification cache en réalité une volonté pure et simple de déréglementation, de dérégulation et, finalement, de « moins d'État ». Comme le souligne le Conseil d'État dans son rapport sur l'inflation législative, le nombre des normes risque de continuer à croître : la « multiplication des sources externes, le droit européen en particulier, en même temps que l'apparition de nouveaux domaines

Qu'avez-vous fait pour maintenir les services publics en milieu rural ou dans les quartiers les plus sensibles ? Qu'avez-vous fait pour renforcer la confiance de nos concitoyens en la parole publique ? En tout cas, il est clair que ce projet de loi ne répondra en rien aux attentes de nos concitoyens. Ce sont les parlementaires, qui sont

Alexis de Tocqueville en 1856, les Français sont plus doués pour la révolution que pour les réformes. Ces propos n'ont rien perdu de leur pertinence, et puisque nous ne pouvons pas faire la révolution tous les quatre matins, nous devons composer avec cette inclination nationale. Cela vaut tout particulièrement pour notre administration, dont l'abondance et la complexité font notre réputation au-delà même de nos frontières. La tentation est grande de faire table rase du passé, de repartir de zéro, mais elle est illusoire. Nous devons donc travailler sur l'existant pour améliorer l'action publique, en gardant à l'esprit ses deux raisons d'être : assurer la permanence de l'organisation sociale et servir l'intérêt général.

mais aussi envers les étrangers, qui aiment notre pays pour la richesse de sa culture et de ses paysages plutôt que pour la complexité de ses règles et de ses formulaires. Ce projet de loi visant à accélérer et à simplifier l'action publique va donc dans le bon sens, mais il est à la révolution ce que le Canada Dry est à l'alcool : ça y ressemble, mais ce n'en est pas

concernant le titre II, transférer des compétences des ministères aux préfets améliorera l'action de l'État. Il s'agit de confier plus de responsabilités aux acteurs de terrain, de faire le pari que l'action publique est plus efficace lorsqu'elle est menée par ceux qui sont en prise directe avec les spécificités locales. Nous avons besoin d'une action publique plus décentralisée et plus déconcentrée, s'exerçant au plus près de nos territoires et de nos concitoyens. Ce sont nos forces vives que nous étouffons en suspendant les destins aux décisions, parfois absconses, souvent obscures, de l'administration française.

certaines d'entre elles ne vont pas assez loin. Ainsi, l'article 26 permet aux entrepreneurs d'anticiper le début de certains travaux de construction sans attendre la délivrance de l'autorisation environnementale, aux frais et risques du demandeur.

cela revient à leur dire : « Prêtez-moi votre montre et je vous dirai l'heure. » Plus fondamentalement, ce texte apportera des aménagements utiles pour nombre de nos concitoyens, mais il échouera à placer l'administration à leur service, et ceux-là resteront dans la dépendance de celle-ci.

Tout d'abord, l'article 34 simplifie les conditions de vente en ligne des médicaments. Censée garantir un meilleur accès aux produits pharmaceutiques, à prix moins élevés, cette évolution de la réglementation a surtout coalisé les pharmaciens contre craignent que la création de plateformes de vente en ligne n'engendre une concurrence dangereuse au détriment des officines les plus petites. Dans les territoires ruraux, les officines créent un véritable lien social. Elles favorisent une dynamique positive des centres-bourgs, qui, aujourd'hui, sont largement délaissés tant par les médecins que par les administrations, les services publics ou les commerces de proximité. De plus, les pharmaciens expriment leur volonté de mieux s'inscrire dans le parcours de soins des patients. Ils font ainsi évoluer leur profession accès à la télémédecine dans les officines, pratique de la vaccination, etc. Ce relais sécurise le malade dans un environnement qui le protège, et nous le soutenons. le dispositif de l'article 34 va à l'encontre des récentes décisions nationales prises pour favoriser le bon usage et la sécurité du médicament en confirmant le rôle de conseil du pharmacien. La commission spéciale a largement amendé cet article, et je m'en réjouis. réjouis. Quant à l'article 43, qui vise à encourager les TPE à mettre en place des dispositifs d'intéressement des salariés au résultat de l'entreprise par une décision unilatérale de l'employeur,

Les salariés des TPE en sont très majoritairement exclus, car ces petites structures entrepreneuriales ne disposent pas des moyens nécessaires en termes de gestion des ressources humaines. C'était une occasion d'y remédier.

J'ai bien noté que ce gouvernement entend aller encore plus loin : un certain nombre de suppressions ont été annoncées lors du quatrième comité interministériel de la transformation publique.

à 120 000 euros au total, dont 100 000 euros pour la seule Commission d'évaluation des politiques publiques de l'État outre-mer. Enfin, il faut souligner que certaines suppressions ne se produiront que sur le papier,

la future loi 3D ou simplement d'utiliser un véhicule législatif opportun ? Là encore, la déconcentration ne se traduira pas par des économies de gestion, puisqu'il s'agit seulement de transférer le pouvoir de décision de l'administration centrale vers les administrations déconcentrées. L'étude d'impact laisse même entrevoir un risque de dérapage budgétaire, certes

Force est de constater, pourtant, que le Gouvernement a une fâcheuse tendance à ne les appliquer que de manière parcellaire. Du point de vue purement formel, il semble impossible de contester la volonté d'accélération de l'exécutif le Sénat a disposé de seulement deux semaines pour examiner un texte qui touche aux secteurs régaliens, à la santé, à l'économie, à la culture et à bien d'autres domaines encore ... Comme pour d'autres débats,

Vous comprenez donc, mes chers collègues, que ce projet de loi dit de « simplification » n'est aucunement d'un abord aisé. L'exercice d'analyse est d'autant plus délicat que ce texte est dépourvu de colonne vertébrale et qu'il s'agit -pardonnez-moi

si elles sont recherchées, c'est, en théorie, pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Mais, concrètement, que signifie une action publique efficace ? En matière de gestion, les Anglo-saxons parleraient d'efficience : il

qu'elles offrent un service public de qualité aux citoyens sur l'ensemble du territoire et qu'elles garantissent le respect et l'effectivité de leurs droits. Sans cette « obligation de résultats » qui incombe à la puissance publique, « accélération » et « simplification » ne sont que de vains mots. Autrement dit, elles ne sauraient constituer ni l'essence ni le but ultime de l'action publique. Ce ne sont pas des objectifs en soi- soi- de même que réformer n'est pas une fin en soi, car on peut très bien réformer pour le pire - ; ce ne sont que des moyens. Malheureusement, trop souvent dans ce texte, l'exécutif semble avoir oublié de lier obligation de moyens à obligation de résultats. Beaucoup de comités ou de commissions sont supprimés, au motif qu'ils seraient inutiles ou que leurs procédures seraient trop lourdes, sans que soit réellement démontré l'impact positif de ces suppressions en termes d'amélioration de l'action publique et de qualité du service public. Au contraire, certains articles peuvent légitimement faire craindre une nette altération, pour ne pas dire une franche détérioration. Sans établir une liste à la Prévert, j'illustrerai mon propos par quelques exemples.

ne proposer qu'un service numérique, sans aucun guichet en préfecture, à une population souvent en situation de vulnérabilité et d'incapacité à accéder au numérique ou à naviguer au sein de la complexité

met en oeuvre des engagements majeurs du Gouvernement, pris notamment lors du dernier comité interministériel de la transformation publique : rapprocher l'administration du citoyen en simplifiant les démarches et faciliter le développement des entreprises en accélérant les procédures administratives.

neuf mois après l'adoption du projet de loi organique réformant le statut d'autonomie de la Polynésie française, sur des déclarations du Gouvernement fortement attendues par les Polynésiens, en supprimant la

qui peuvent nourrir des tensions inutiles entre les Polynésiens et l'État. Notre groupe a déposé un amendement de suppression de cet article, afin de préserver le lien nécessaire garanti par cette structure. ! L'article 33 traite de l'épineux problème de l'ONF. Les dispositions proposées sont des mesures de fond qui, si elles étaient mises en oeuvre, transformeraient le fonctionnement, le statut du personnel et l'objet même de l'ONF. Elles dépassent très largement le cadre de l'établissement public pour ce qui concerne l'exécution de missions de police judiciaire par des salariés de droit privé,

dès lors, pas opportun, les implications juridiques pouvant être lourdes. Concernant la gouvernance de cet établissement, nous nous inscrivons dans la droite ligne de la résolution du Congrès des maires, qui appelle à ce que son évolution soit envisagée en concertation approfondie avec les élus.

Enfin, l'article 36 prolonge et complète l'habilitation issue de l'article 50 de la loi Essoc, dans la perspective d'une réforme de l'ensemble des modes d'accueil et de pilotage local. J'insisterai sur le fait

En tout état de cause, il n'est pas question que les normes retenues aboutissent à la fermeture de places d'accueil existantes. Il faut conclure, mon cher collègue ! De même, le schéma départemental des services aux être transformé en outil de planification obligatoire de l'offre. Il faut laisser toute sa place à la négociation, dans le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales et sans dilution de la place des élus, afin de préserver une approche au plus près des territoires.

premier lieu, pourquoi nous imposer d'examiner ce texte à marche forcée ? Y avait-il urgence à prendre des mesures concernant l'archéologie préventive ?

au fait que le Gouvernement nous présente ce texte comme une des résultantes des consultations effectuées dans le cadre du grand débat national de l'an dernier.

que de l'utilité de la commission consultative des baux ruraux, de l'opportunité de conserver la Commission centrale des évaluations foncières ou de la pertinence de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

Ainsi, en pleine réflexion sur les restitutions- on sait le travail accompli sur le sujet par la commission de la culture du Sénat et sa présidente, Catherine Morin-Desailly -, vous entendiez supprimer la Commission scientifique nationale des collections. Nous sommes nombreux à le regretter. Au-delà, le besoin de transformation, de simplification et d'accompagnement de l'action publique relève d'une préoccupation pérenne des responsables politiques et d'une attente de nos concitoyens. J'en arrive ainsi à mon troisième motif d'étonnement, nourri par le décalage entre l'ambition politique affichée au travers de ce texte et son contenu. Nos concitoyens ont besoin de présence et d'échanges efficaces avec les services déconcentrés de l'État.

qu'évoquait déjà, en 1969, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas ? Les dispositions de ce projet de loi sont avant tout issues d'une administration qui se parle à elle-même. Elles ne vont donc pas suffisamment loin pour que la simplification infuse dans la vie de nos concitoyens, parce qu'elles ont pour point de départ l'administration elle-même et non le parcours de l'administré. Mon quatrième motif d'étonnement, enfin, tient à ce que ce projet de loi révèle de la cohérence de l'action gouvernementale et de son calendrier. Pour que cohérence il y ait, n'aurait-il pas fallu mener une réflexion sur le périmètre de l'État et sur l'application du principe de subsidiarité ? Quelle peut être la cohérence de ce texte quand les consultations sont en cours afin de finaliser le projet de loi 3D, porté par la ministre de la cohésion des territoires texte en constitue-t-il un premier volet ou s'agit-il d'une initiative connexe ? Nous n'en savons rien. Faute de ligne directrice, ce projet de loi s'apparente à un inventaire à la Prévert. Il est composé de dispositions plus ou moins opportunes, plus ou moins bien préparées, plus ou moins bien acceptées par les acteurs. De surcroît, en cherchant à faire du chiffre, vous avez pris le risque d'inquiéter certaines professions. Ce n'est, en effet, pas au détour d'un texte de cette nature que l'on réforme l'économie de la distribution du médicament et le maillage du territoire par les officines, les missions et l'organisation de l'ONF ou encore la place des assurances dans les procédures de fixation des honoraires des avocats. Ce texte fourre-tout ne peut être le véhicule de réformes de fond qui méritent études, concertation et débats approfondis. Néanmoins, certaines

la simplification ne doit pas seulement être rhétorique ; elle doit se traduire concrètement pour nos concitoyens et nos entreprises. À ce titre, le projet de loi va dans le bon sens en simplifiant l'administration et certaines démarches

encore, comme cela a déjà été dit, l'administration s'est trop souvent révélée incapable de fournir les informations demandées, notamment sur les dispositions des ordonnances pour lesquelles une habilitation est demandée par le Gouvernement. Quelle est la première victime de la marche forcée imposée par le Gouvernement ? La démocratie parlementaire, sans parler de l'atteinte aux principes de sécurité juridique, de clarté du droit et de sincérité des débats

l'article permettant la suppression de la Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux (CCPNBR). Les commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux interviennent dans le domaine du statut du fermage, notamment pour proposer aux autorités administratives compétentes les minima et les maxima qui servent au calcul du prix du fermage. En cas de carence de ces commissions, la charge de formuler ces propositions revient à la Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. celle-ci a été de moins en moins sollicitée, puisqu'elle ne conserve, en réalité, qu'un rôle supplétif de celui des commissions départementales et qu'il revient, dans tous les cas, au préfet du département de procéder lui-même à la fixation des minima et des maxima.

souhaitable. Cette commission propose les minima et les maximaqui encadrent les loyers des baux ruraux. Pour ce faire, elle réunit notamment des représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers, des syndicats agricoles et des chambres d'agriculture. Elle ne joue qu'un rôle subsidiaire par rapport aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, puisqu'elle n'intervient que dans l'hypothèse où ces dernières ne seraient pas parvenues à un accord. La supprimer reviendrait en réalité à permettre à l'État de fixer les minima et les maxima précités sans même rechercher l'accord des premiers concernés. Dans un contexte de raréfaction du foncier, de nature à renforcer localement les situations de conflit, il est préférable de maintenir une instance nationale de concertation, qui peut jouer un utile rôle de garde-fous en cas de dysfonctionnement des commissions départementales, plusieurs organismes professionnels siégeant à la CCPNBR. Par ailleurs, le 6 février dernier, le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, a indiqué devant le Sénat que le Gouvernement travaillait au projet de loi foncière.

qu'il est proposé d'opérer est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, la disposition législative qui serait supprimée ne vise pas expressément la commission départementale de la gestion de l'espace, comme indiqué dans l'objet de l'amendement, mais le principe de la consultation d'une commission associant les professionnels dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de gestion de l'espace rural. Or on peut vouloir conserver dans le code ce principe d'une consultation des professionnels. Par ailleurs, si une évolution doit intervenir, c'est plutôt dans le cadre de la réforme globale qu'opérera le projet de loi foncière déjà évoqué. Pour autant, compte tenu de la nécessité de faire évoluer notre droit, je propose au Sénat de suivre l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

été supprimée de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime par l'article 2 du décret du 7 août 2017 portant mise à jour des livres I et II de la partie réglementaire de ce code, le toilettage proposé par le sénateur Gremillet nous paraît tout à fait opportun.

ces comités donnent un avis sur les autorisations d'aménagement accordées par les bailleurs aux preneurs de terres agricoles. Il s'agit d'instances spécialisées, mobilisant peu d'acteurs : le préfet et cinq représentants des professionnels agricoles. comités interviennent dans une phase précontentieuse, en réglant les différends entre bailleurs et preneurs sur les travaux à réaliser, avant une éventuelle saisine des tribunaux paritaires des baux ruraux. à la suppression à la suppression de ces comités à l'occasion de l'examen par la commission des affaires économiques d'une proposition de loi relative à l'accaparement des terres et au développement du biocontrôle, en 2017.

Par exemple, j'ai proposé que l'on se penche sur les missions très similaires du Conseil national de l'alimentation et de l'Observatoire de l'alimentation, coûtant respectivement 408 000 et 450 000 euros par an ; des synergies peuvent être trouvées, me semble-t-il.

De plus, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire aurait pu, le cas échéant, reprendre les missions de cette commission. Nos concitoyens attendent de la rationalité dans la gestion des deniers publics ; ils souhaitent que chaque euro dépensé le soit à bon escient.

fois entre 2012 et 2017. Dans son rapport d'avril 2018, elle a mis en lumière, au moyen de données statistiques, une surpopulation carcérale, particulièrement criante au sein des maisons d'arrêt. concluait ainsi : « Il appartient désormais aux différents acteurs de se saisir de cette question, en veillant à ce que le placement en détention soit l'exception et en préférant des mesures alternatives à l'emprisonnement. » La commission constatait les difficultés liées à un manque important d'effectifs et de moyens et plaidait pour que la question de la surpopulation carcérale soit placée au centre des préoccupations de tous les acteurs de la politique pénale. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 30 janvier dernier, a condamné la France pour les conditions de détention dans ses prisons surpeuplées. de prendre des mesures pour résorber la surpopulation carcérale. Il se trouve que l'une des explications de la surpopulation carcérale tient au recours massif à la détention provisoire.

permettant la résorption définitive de la surpopulation carcérale. Cette énième condamnation ne vise pas une personne, mais plus globalement un système carcéral, a affirmé lors d'une conférence de presse Nicolas Ferran, le référent des contentieux à l'Observatoire international des prisons (OIP).

Outre ces recommandations, la justice européenne a condamné la France à payer près de 500 000 euros aux détenus concernés. Dans ce contexte, notre pays se donne pour objectif de construire toujours plus de prisons, sans réfléchir

à la décroissance carcérale ; la détention provisoire est la clé de voûte de cette réflexion. Comment l'encadrer plus strictement ? Pour répondre à cette question, la Commission de suivi de la détention provisoire devrait,

déplorait l'incapacité de l'appareil statistique à appréhender le phénomène de la détention provisoire, ainsi qu'une dégradation de la lisibilité des données. Son président avait déclaré en 2017 que la chancellerie ne prêtait plus attention à ce sujet depuis quelques années. Pour ces raisons,

Ces deux amendements identiques sont contraires à la position de la commission spéciale. Ils tendent à supprimer l'article 2 du projet de loi, qui supprime la Commission de suivi de la détention provisoire. conduirait au maintien d'une commission dont le mandat des membres est arrivé à expiration en avril 2018, sans renouvellement à ce jour, et qui n'a plus aucune activité depuis presque deux ans. En outre, la commission en question ne produisait pas elle-même de données statistiques sur la détention provisoire, et ses missions semblent pouvoir être assurées par le ministère de la justice, dans le cadre de l'évaluation du recours à la détention provisoire.

La suppression du Conseil national de l'aide aux victimes (CNAV) apparaît aujourd'hui comme une volte-face du Gouvernement. En effet, après avoir annoncé, à l'occasion de l'adoption de la loi du 3 août

l'exécutif considère aujourd'hui que ses missions pourraient être directement exercées par le ministère de la justice. On évoque notamment la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes et le Comité interministériel de l'aide aux victimes, dont la dernière réunion s'est tenue en mars 2019. Cependant ce comité interministériel, composé de membres du Gouvernement, ne saurait remplacer le Conseil national de l'aide aux victimes, qui réunissait des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide aux victimes, des personnalités qualifiées et le directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ainsi que des parlementaires. Le CNAV est chargé de coordonner l'action du Gouvernement avec celle des autres instances, non gouvernementales, pour garantir et renforcer le droit des victimes. L'existence de ce comité témoigne que la politique publique d'aide aux victimes est un élément majeur de la politique pénale. Durant le quinquennat précédent, la garde des sceaux l'avait réuni plusieurs fois, rappelant les enjeux liés à l'amélioration de la prise en charge des victimes et la nécessité de dessiner avec les associations de nouvelles perspectives en matière d'accompagnement et d'indemnisation. On peut effectivement s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce conseil n'a pas été réuni ces dernières années,

En outre, il apparaît que les missions du CNAV peuvent être exercées par la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, qui coordonne l'action des différents ministères en matière de suivi et d'accompagnement des victimes et travaille en partenariat avec des associations oeuvrant dans ce domaine et différents acteurs locaux.

secrétaire d'État. Il s'agit de rétablir l'article 4, qui supprime l'Observatoire de la récidive et de la désistance. Chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et la réitération,

notamment ceux de l'administration pénitentiaire et de la direction des affaires criminelles et des grâces, afin de produire les analyses qui permettront, conformément aux objectifs du Gouvernement figurant dans la loi de programmation du 23 mars 2019, d'améliorer la lutte contre la récidive.

De plus, pour suivre plus facilement le parcours des condamnés et examiner si ces derniers récidivent ou non, la loi du 23 mars 2019 a modifié un article du code de procédure pénale relatif au traitement Cassiopée, qui comporte les données de toutes les procédures pénales suivies dans les juridictions, nous fournissant ainsi un autre éclairage statistique. Il est désormais prévu que les données nominatives figurant dans ce traitement puissent être exploitées à des fins statistiques. Ainsi, avec la mobilisation des services

la désistance semble encore en activité, ainsi qu'en témoigne l'organisation d'un colloque dans les locaux de l'Assemblée nationale en juin dernier. Par ailleurs, il convient de constater la plus-value apportée par l'analyse pluridisciplinaire des données récoltées par cet observatoire permet de dégager de véritables axes de réflexion en la matière. Les missions de cet observatoire auraient pu être exercées par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, chargé d'étudier les évolutions statistiques en matière de délinquance au sein de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, mais le Gouvernement a récemment émis le souhait